Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici réunis pour examiner le texte adopté par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur la proposition de loi visant à permettre l'implantation de panneaux photovoltaïques sur des friches.

présente proposition de loi a été déposée par Didier Mandelli et plusieurs de ses collègues dans l'objectif de faire enfin aboutir ce dispositif consensuel et équilibré, qui répond à une demande formulée de longue date par les élus du littoral. loi Littoral, freine actuellement le déploiement de l'énergie photovoltaïque dans de nombreuses communes littorales. En effet, en application du code de l'urbanisme, « l'extension de l'urbanisation », c'est-à-dire les constructions nouvelles, n'est autorisée sur le territoire de ces communes qu'à proximité des « agglomérations et villages existants ». Si des dérogations à ce principe ont été définies par le législateur, notamment pour les cultures marines et les activités agricoles et forestières, aucune dérogation n'est prévue à ce jour pour les installations nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil. En outre, En outre, le juge administratif rappelle, dans une jurisprudence constante, qu'il considère les installations photovoltaïques comme une « extension de l'urbanisation » qui n'est permise, sur le territoire des communes littorales, qu'en continuité avec les constructions existantes. De nombreuses communes littorales souhaitant installer des panneaux solaires à distance des habitations, afin de favoriser leur acceptabilité sociale, se trouvent donc dans une impasse juridique. Tel est le cas de la commune de L'Île-d'Yeu, dans laquelle je me suis rendue le 3 février dernier avec Didier Mandelli : elle porte depuis près de dix ans un projet de parc photovoltaïque qui permettrait d'accroître son autonomie énergétique. L'implantation de ce parc est envisagée dans une ancienne décharge, afin de ne pas empiéter sur des surfaces naturelles. Le projet se heurte toutefois à des freins juridiques, notamment du fait de la loi Littoral. À l'heure où la France affirme ses ambitions en matière de transition énergétique, cette situation, que connaissent de nombreux territoires, n'est pas satisfaisante. Rappelons que la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte a prévu de porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans notre production d'électricité d'ici à 2030. Par ailleurs, la loi Climat et résilience a prévu la déclinaison de ces objectifs à l'échelle régionale, afin d'ancrer la transition énergétique au niveau local.

Cette problématique est accentuée dans les régions insulaires, souvent fortement dépendantes d'énergies fossiles importées du continent, dont l'approvisionnement peut être instable et le coût élevé. À cette difficulté s'ajoutent des contraintes urbanistiques fortes liées à la géographie des îles : les communes littorales s'y étendent parfois loin dans les terres et à distance du rivage, en particulier dans les outre-mer. Conscient de la nécessité d'un assouplissement de la loi, dès 2015, le législateur a autorisé l'implantation d'éoliennes à distance des villes et villages en zone littorale, en métropole comme en outre-mer. L'article unique de cette proposition de loi vise à étendre cette possibilité aux installations photovoltaïques. Afin de ne pas accroître l'occupation des sols, il est toutefois prévu que cette dérogation ne s'applique qu'à des friches, c'est-à-dire à des sites qui ne sont plus exploités, dont la liste sera fixée par décret. Cette dérogation est encadrée de manière stricte afin de garantir la protection des milieux littoraux d'une part, les projets seront autorisés au cas par cas par l'autorité compétente de l'État, sur la base d'une étude d'incidence démontrant notamment que le projet ne porte pas atteinte à l'environnement ou aux paysages ; d'autre part, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sera consultée avant toute autorisation. En commission, nous avons encore renforcé les garde-fous, en prévoyant la consultation du Conservatoire du littoral pour l'établissement de la liste des friches concernées et en précisant le champ de l'étude d'incidence environnementale qui sera remise par le maître d'ouvrage. Le recensement des friches n'a pas encore débuté, mais une vingtaine de sites pourraient être concernés. Vous l'aurez compris, notre commission approuve pleinement ce dispositif qui aidera les communes littorales à s'engager dans une démarche de transition écologique et à participer à l'effort collectif en faveur des énergies renouvelables. J'ai conscience que l'objet de ce texte est très circonscrit et que certains d'entre vous, mes chers collègues, auraient souhaité aller plus loin pour favoriser le déploiement des activités favorables à la transition écologique en zone littorale. Je pense toutefois que nous devons considérer ce texte comme une première étape dont nous pouvons nous satisfaire aujourd'hui. Il importe à présent que cette proposition de loi aille au terme de la navette parlementaire. Malheureusement, ce texte ne sera pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avant la suspension des travaux parlementaires. Je le regrette d'autant plus que cette proposition de loi satisfait à la fois le Gouvernement, les députés et les acteurs de terrain son adoption définitive par le Parlement d'ici à la fin du mois aurait donc probablement été une simple formalité. Même si le calendrier parlementaire est très contraint en cette fin de législature, il me semble qu'un examen « éclair

En tout état de cause, on peut espérer que la prochaine législature nous permette enfin d'aboutir sur ce sujet et de concrétiser l'évolution de bon sens que nous proposons. Vous l'aurez compris, madame la secrétaire d'État, il s'agit de mettre nos actes en cohérence avec nos ambitions en matière de transition énergétique et de permettre à l'énergie photovoltaïque de trouver sa place dans les communes littorales. La parole est à Mme la secrétaire

essentiels de notre nouveau mix énergétique : la sobriété, les énergies renouvelables et le nucléaire. Nous devons développer cette ambition, en particulier autour de l'énergie photovoltaïque,

ont déjà été déposés. Les mesures adoptées ces dernières années portent leurs fruits, avec un niveau record de raccordement de plus de 2 gigawatts l'an dernier,

pour identifier toutes les friches susceptibles d'accueillir des projets photovoltaïques. Cette étude est désormais finalisée. Je suis très heureuse de vous annoncer que la liste des 874 sites potentiels,

En cohérence totale avec l'enjeu de mobiliser des friches pour les projets photovoltaïques, la présente proposition de loi vise à permettre d'installer des dispositifs de production d'électricité photovoltaïque sur des friches localisées dans les zones soumises à la loi Littoral.

avec celle que nous menons, du local au national. Elle allie développement des énergies renouvelables et mobilisation des espaces les mieux adaptés, là où les enjeux environnementaux sont les plus limités. C'est dans cet esprit aussi que nous encourageons l'installation de panneaux solaires sur les toitures, en facilitant l'accès au tarif de rachat de l'électricité produite. Notre priorité en matière de friches est leur valorisation, qui permet d'économiser du foncier et de lutter contre l'artificialisation des sols. C'est dans cette optique que nous encourageons leur reconversion.

en prévoyant que ces installations ne pourront être permises qu'à titre exceptionnel, par l'autorité compétente de l'État et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Je suis évidemment, tout comme vous, particulièrement attachée à ce que ce texte limite la dérogation aux cas où le projet photovoltaïque satisfait mieux l'intérêt public qu'un projet de renaturation. Il faut que nous sachions vraiment construire ensemble ces

le groupe RDPI soutient pleinement cette initiative de Didier Mandelli et plusieurs de ses collègues en faveur de l'implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites jugés dégradés- en l'occurrence, des friches.

L'article unique présenté en commission, amendé trois fois et dont nous débattons aujourd'hui en séance publique, vient donc confirmer la volonté du législateur, avec un véhicule législatif cette Depuis 1986, comme cela a été rappelé, les constructions nouvelles dans les communes littorales ne peuvent être réalisées qu'en continuité avec les « agglomérations et villages existants », en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. de l'urbanisme. La jurisprudence administrative est claire et constante sur ce point : l'implantation de parcs photovoltaïques est concernée, elle n'est donc permise qu'à cette condition. Des dérogations au principe général ont pourtant déjà été prévues. C'est notamment le cas pour les cultures marines et pour les activités agricoles et forestières. Depuis 2015, c'est aussi le cas pour l'édification d'éoliennes. La justification est l'existence possible de nuisances, notamment sonores, pour les riverains,

totalement dépendantes des énergies fossiles. À plusieurs endroits du territoire, en métropole et outre-mer, un conflit existe entre la norme édictée il y a bientôt quarante ans et les objectifs actuels fixés par la France en matière de transition énergétique. Au regard des défis environnementaux que nous devons relever, cette dérogation à la loi Littoral représenterait une avancée souhaitable et légitime. Ainsi, à Fouesnant, dans le Finistère, un projet d'implantation de parc solaire sur une ancienne décharge ne peut pas voir le jour, alors même que la terre ne peut pas être rendue à l'agriculture.

Pour ce qu'elle représente, dans son bilan et sa valeur protectrice, nos élus sont très attachés à la loi Littoral, mais celle-ci doit aussi être adaptée aux nouveaux enjeux, qui sont multiples et transverses : autonomie énergétique, densification urbaine, agriculture, ou encore accès aux services numériques. Littoral est aujourd'hui perçue comme un cadre trop rigide, interprété de manière restrictive par le juge administratif. Elle a freiné le bétonnage de nos côtes ; nous nous en félicitons. Mais elle génère également incompréhensions et tensions au niveau local.

Je pense à la question de la desserte numérique en zone littorale : on pourrait ouvrir la possibilité d'implanter des antennes en discontinuité de l'urbanisation. Je pense aussi à la question agricole : comment justifier qu'un exploitant soit entravé dans son développement lorsqu'il souhaite implanter son logement à proximité de son exploitation ? Je pense enfin à la densification de nos villages littoraux, qui nécessiterait de permettre les constructions dans les dents creuses.

il a été rappelé lors de nos discussions, il y a urgence sur nos territoires soumis à la loi Littoral, qui sont confrontés à certains obstacles, même si le but de cette loi est de préserver ici prévue au principe de l'extension de l'urbanisation de l'aménagement du littoral est acceptable, car elle est strictement encadrée et maîtrisée. La contrainte à laquelle nous sommes soumis tient au fait que notre pays doit déployer intelligemment et avec ambition des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, tout en préservant les terres agricoles et les espaces naturels. Il faut donc trouver des solutions intermédiaires, comme l'utilisation de friches, si l'on veut limiter l'artificialisation des sols. Notre groupe s'est largement investi afin de freiner ce phénomène tout en trouvant des solutions équilibrées entre territoires. Cette proposition de loi répond à cette double évolution au sein même des territoires du littoral. Sous certaines conditions, nous pourrons installer des panneaux solaires sur des friches préalablement identifiées. Je connais l'engagement du Gouvernement en ce sens. L'enjeu est important et représente plusieurs gigawatts de capacités. Ainsi, en installant du photovoltaïque sur des sites dégradés, on peut concourir aux objectifs français de déploiement des énergies renouvelables et de neutralité carbone d'ici à 2050 tout en préservant nos sols. Je crois profondément à l'usage de panneaux solaires sur des sols ayant une activité principale différente. Ainsi, pas plus tard qu'hier, j'organisais une visite sur mon territoire, dans la région toulousaine, à la rencontre d'un acteur local qui défend un projet très ambitieux Là encore, il s'agit de produire des énergies renouvelables sur des sols qui continueront à être cultivés. Pour l'heure, certains obstacles administratifs doivent être levés ; nous devons également définir un cadre juridique pour l'agrivoltaïsme. Dans nos régions où l'agriculture est fortement impactée par le réchauffement climatique, l'agrivoltaïsme est synonyme d'espoir pour notre mix énergétique, pour la préservation de nos terres agricoles et pour un revenu complémentaire garanti à nos agriculteurs. J'ai l'habitude de le dire dans cet hémicycle, mais je veux le répéter une nouvelle fois : l'ambition, l'innovation, la recherche et des moyens adéquats sont les clés de nos futures révolutions énergétiques et agricoles. Cette proposition de loi s'inscrit tout à fait dans cette démarche en ce qu'elle propose une adaptation de la réglementation de certaines zones à nos besoins énergétiques. L'étude d'incidence, qui conditionne l'installation de panneaux solaires sur une friche, est la garantie d'un projet équilibré pour le territoire où il prend place. Il sera le meilleur choix lorsque la renaturation du site ne sera pas possible il n'aura pas d'impact sur la salubrité ou la sécurité publique. Enfin, il contribuera à la protection de notre environnement et de notre biodiversité, tout en respectant les paysages de nos littoraux. C'est certainement cet outil qui fait que cette adaptation souhaitée est acceptable et qu'elle remplira ses objectifs sans effets négatifs sur nos paysages. Je terminerai mon propos en soulignant la modification du texte qui donne une place particulière au Conservatoire du littoral dans l'établissement de la liste des friches sur lesquelles pourront être autorisés les projets photovoltaïques. En tant qu'élu au conseil d'administration de cet organisme, et connaissant la qualité du travail qui y est fourni, je ne peux que me satisfaire de son implication. Le mécanisme proposé par ce texte a été longuement discuté et a déjà fait l'objet d'un accord avec l'Assemblée nationale. J'ai exposé les raisons pour lesquelles il est solide, justifié et apporte de la flexibilité à la loi Littoral.

sur le site d'un ancien centre d'enfouissement technique. Ce projet est censé occuper une surface de 1,5 hectare sur les 5 hectares du site et permettre, grâce à l'ensoleillement dont bénéficie l'île, et la Vendée en général, de gagner en autonomie énergétique, pour arriver à 35 % des besoins. Le projet se heurte à des obstacles juridiques relatifs à la loi Littoral, qui encadre les conditions d'aménagement et d'occupation des sols dans les quelque 1 200 communes littorales françaises. Selon la loi, à laquelle nous sommes tous très attachés, les installations photovoltaïques doivent être considérées comme une « extension de l'urbanisation ». L'implantation de parcs photovoltaïques n'est donc permise sur le territoire des communes littorales qu'en continuité des constructions existantes. J'avais alerté, dès 2017, le Gouvernement sur cette situation, qui m'a immédiatement semblé être à contre-courant des objectifs que nous nous fixons en matière de réduction de nos émissions de CO2 et de notre dépendance aux énergies fossiles. Cela fait plus de dix ans que le maire de L'Île-d'Yeu, Bruno Noury, ne parvient pas à concrétiser ce projet, à l'instar d'autres élus du littoral qui aspirent à développer une énergie décarbonée sur leur territoire.

Ce texte est donc le fruit d'un long cheminement, comme je l'ai rappelé en commission. Le sujet a déjà été abordé dans la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte, dans la loi pour l'économie bleue, dans la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux de notre ancien collègue Michel Vaspart, et enfin, plus récemment, dans la loi Climat et résilience. Il aura fallu attendre Il aura fallu attendre cette dernière pour que nous puissions nous accorder sur cette mesure essentielle pour nos élus du littoral. Le Conseil constitutionnel a pourtant jugé que cette mesure représentait un cavalier législatif dans la loi Climat. Ainsi, selon lui, on ne pouvait pas faire de lien entre l'installation de panneaux photovoltaïques et l'objectif de ce texte. Vous me permettrez à ce stade de vous faire part de mon incompréhension face à cette décision. Je me réjouis que nous puissions examiner aujourd'hui cette proposition de loi, juste avant la suspension de séance imposée par les échéances électorales, et je remercie le rapporteur, Jean-Claude Anglars, autant de la qualité de son travail que d'être venu en Vendée.

La proposition de loi a fait l'objet d'une mesure d'examen particulière en commission, laquelle l'a votée à l'unanimité, ce dont je me félicite, puisque cela confirme qu'il s'agit bel et bien d'une mesure de bon sens. Je remercie également le

lors de l'examen de la loi Climat et résilience, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires (GEST) avait soutenu le dispositif que nous examinons aujourd'hui, tout en étant très attentif à la dérogation portée à la loi Littoral, toute dérogation à celle-ci nécessitant d'être scrupuleusement pesée et évaluée. Vous connaissez notre vigilance sur le sujet. À l'époque, le travail en commission mixte paritaire avait permis de strictement limiter la dérogation à la loi Littoral, en introduisant une série de garanties, en prévoyant que les autorisations d'implantation soient accordées à titre exceptionnel, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, et avec une étude d'incidence pour s'assurer que les enjeux de protection de l'environnement soient bien pris en compte. Enfin, la dérogation à la loi Littoral n'était possible que si le projet d'implantation de panneaux photovoltaïques s'avérait plus bénéfique qu'une opération de renaturation,

pour que l'étude d'incidence démontre bien que le projet d'implantation de panneaux photovoltaïques sur les friches n'est pas de nature à porter atteinte à la biodiversité, qui peut être importante sur ces territoires. Je crois que cela répond, madame la secrétaire d'État, à la préoccupation que vous venez d'exprimer. Un second garde-fou a été utilement ajouté : la consultation préalable du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur le décret fixant la liste des friches éligibles au dispositif. Ce texte permettra donc aux collectivités littorales porteuses de projets d'implantation de panneaux photovoltaïques de sortir de l'impasse juridique, avec un encadrement qui nous semble suffisamment protecteur. Cette proposition de loi mise clairement sur le photovoltaïque pour augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité française, mais son impact sera néanmoins limité, il faut le dire, car seulement une vingtaine de sites seraient concernés par le dispositif. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous accusons un énorme retard dans le développement des énergies renouvelables en France. Un récent classement de l'institut de statistiques européen Eurostat révèle que la France est le seul pays européen à avoir manqué son objectif de 23 % d'utilisation du renouvelable dans sa consommation finale d'énergie en 2020. Alors que

nécessaire une accélération du déploiement des énergies renouvelables. M. le rapporteur a appelé voilà quelques instants à faire preuve de volontarisme dans ce domaine,

peu onéreux et facile à installer, qui est la principale solution technologique à notre portée, y compris financièrement : c'est de loin le retour sur investissement le plus rapide. Je vous cite encore, monsieur le rapporteur-

probablement la seule pour que la France renforce son indépendance énergétique. Il s'agit d'un enjeu central, qui relève de la responsabilité politique de la représentation nationale, tout particulièrement dans cette période de grande tension internationale.

panneaux photovoltaïques sur des sites jugés dégradés en zone littorale. La disposition alors adoptée avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Tout d'abord, reconnaissons que la problématique de l'adaptation de la loi Littoral à la réalité des territoires pour asseoir leur développement est récurrente au sein de cet hémicycle.

Trop souvent, la loi Littoral a été remise en cause pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, il est question d'autoriser l'implantation de panneaux photovoltaïques dans les friches, y compris si celles-ci ne se trouvent pas en situation de continuité urbaine. Cette dérogation ne serait pas laissée à la main des élus locaux : elle serait autorisée par le préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et encadrée par une étude d'incidence permettant de démontrer que le projet répond bien à plusieurs exigences. Par ailleurs, la liste des friches dans lesquelles ces autorisations pourraient être délivrées serait fixée par décret. Selon le ministère de la transition écologique, ce dispositif concernerait une vingtaine de sites. En commission, le texte a connu des évolutions que nous jugeons favorables. Ainsi, le champ de l'étude d'incidence est étendu aux atteintes à la biodiversité, et n'est plus limité aux seules atteintes environnementales. La liste des friches concernées devra par ailleurs être établie après consultation du Conservatoire du littoral. Ces consultations Ces consultations nous semblent utiles, mais nous regrettons cependant que l'avis des maires et des EPCI concernés ne soit pas prévu. Il s'agit clairement d'une lacune. Sur l'intérêt de cette dérogation à la loi Littoral, nous considérons que l'enjeu de développement de l'énergie solaire dans notre mix énergétique doit être défendu, en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Actuellement, ces installations sont interdites dans la bande littorale de 100 mètres, puisqu'elles ne constituent pas des installations liées à un service public ou à une activité économique qui exige la proximité immédiate de l'eau. Dans les autres parties du territoire communal, les parcs photovoltaïques sont soumis au principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Comme l'ont rappelé les travaux de la commission, la jurisprudence est à ce propos d'une grande constance. La cour administrative d'appel de Marseille vient encore de la confirmer en annulant le permis de construire délivré par le préfet de l'Aude pour le parc photovoltaïque de la société Soleil participatif du Narbonnais, le 9 mars 2021. Une évolution de la loi Littoral sur ce point, de manière très encadrée, comme c'est le cas avec cette proposition de loi est donc la bienvenue pour permettre, par exemple, l'implantation de parcs photovoltaïques au sol sur des sites impropres à l'activité agricole, comme des anciennes carrières ou décharges.

carrières, les gravières ou les centres de stockage des déchets inertes. Cette règle de priorité doit absolument être respectée et l'implantation en zone littorale doit ainsi conserver un caractère purement exceptionnel.

de « réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie par la production énergétique à partir de sources renouvelables », conformément aux textes réglementaires. il importe, même si tel n'est pas le sujet de cette proposition de loi, de réfléchir au développement des énergies renouvelables afin de les placer sous entière maîtrise publique- aujourd'hui, il s'agit d'un secteur très morcelé -, et d'obtenir un véritable plan national de développement et d'aménagement du territoire. Sous réserve de ces observations, nous voterons en faveur de cette proposition de loi. La parole Madame la présidente, monsieur le ministre,

littorales. La loi du 3 janvier 1986, dite loi Littoral, encadre strictement les conditions d'aménagement et d'occupation des sols dans nos 1 200 communes littorales françaises. Si cette loi répond à un objectif louable, celui de concilier développement de l'urbanisme et préservation de l'environnement, elle entrave cependant le développement de l'énergie solaire, puisqu'aucune dérogation n'est effectivement prévue pour les panneaux photovoltaïques. Ce texte, dont je salue les auteurs, vise donc à permettre l'implantation de ces panneaux sur des sites jugés dégradés, et plus particulièrement des friches. C'est aussi un élément du grand puzzle mondial de la lutte contre le réchauffement climatique. La France entamera bientôt son troisième mois à la présidence du Conseil de l'Union européenne, et il est crucial de montrer l'exemple à cet égard en accordant un soutien sans faille à toutes les énergies renouvelables. Nos territoires étant les premiers à le demander, donnons donc à l'échelon local les moyens d'être vecteur d'une transition énergétique nationale et internationale. Je pense notamment à nos collectivités insulaires, dépendantes elles aussi des énergies fossiles. Est-il encore nécessaire de rappeler ici que la consommation d'énergies fossiles est la principale cause des dérèglements climatiques, sans compter les conséquences de certains désastres écologiques conjoncturels comme les marées noires, les fuites des installations offshore ou parfois même leur explosion ? pense ici à l'explosion en 2010 de la plateforme Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique- une plateforme au nom prédestiné, puisqu'elle a fini à 1 500 mètres de fond -, qui a fait onze morts et souillé 2 000 kilomètres de côtes américaines avec 678 000 tonnes de brut libérées dans la nature. Le chiffre astronomique, mais probablement insuffisant, du dédommagement, à hauteur de 21 milliards de dollars, démontre, s'il en était encore besoin, la soif d'énergie à tout prix des pays développés. Une soif d'or noir qui ne diminue pas et qui est aujourd'hui boostée par la demande des pays émergents. Cette compétition pour les ressources fossiles est aussi une source de tensions internationales et, potentiellement, de conflits. Bref, nous avons tout à gagner à soutenir les énergies renouvelables ou plutôt, devrais-je dire, nous avons tout à perdre à ne pas le faire. Cette proposition de loi est donc une évidence et certains, dont je suis, auraient d'ailleurs aimé aller encore plus loin. J'aurais par exemple souhaité pouvoir ajouter à ce texte une mesure permettant l'installation de panneaux photovoltaïques le long des routes et le long des autoroutes.

Positivons cependant en considérant que cette proposition de loi est un premier pas vers plus de souplesse, à terme, sur tous nos territoires, pour une meilleure intégration des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Notre collègue Annick Billon se réjouit de l'initiative des parlementaires, et de Didier Mandelli, en particulier, car elle ouvre une nouvelle perspective à un projet, qu'elle a défendu au ministère de l'écologie avec le maire de L'Île-d'Yeu,

le groupe Union Centriste votera cette proposition de loi, qui reprend une mesure de la loi Climat du 22 août 2021, une mesure adoptée par les deux assemblées avant d'être censurée par le Conseil constitutionnel. Rappelons que les débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle à propos de l'hydrogène, de l'éolien, de la biomasse ou encore du nucléaire ont souvent donné lieu à d'importants désaccords. nous avançons à petits pas, conscients qu'il y a non pas une solution miracle, mais plutôt, comme nous le disions avec Jean-Louis Borloo lors du Grenelle de l'environnement, un bouquet de solutions pour remplacer à terme l'énergie fossile.

d'honneur d'une délégation parlementaire du Grand Khoural de Mongolie, conduite par le président du groupe d'amitié Mongolie-France, M. Chinburen Jigjidsuren. La délégation est accompagnée par notre collègue Philippe Mouiller, qui préside le groupe d'amitié France-Mongolie. Cette visite s'inscrit dans le prolongement du récent déplacement d'une délégation du groupe d'amitié en Mongolie, en septembre dernier, auquel j'ai eu l'honneur de participer. Nous avions reçu un accueil chaleureux de M. Chinburen et du général Sergelen Tsedev, qui l'accompagne aujourd'hui. Cette visite est Cette visite est l'occasion de renforcer encore nos liens, d'identifier de nouveaux champs de coopération interparlementaire. Elle permettra aussi de nouer des contacts économiques avec des entreprises françaises, en particulier dans les domaines de la sécurité civile et des transports.

Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à la délégation du Grand Khoural la plus cordiale bienvenue et un fructueux séjour. Je me permets enfin de saluer la présence de l'ambassadrice de Mongolie en France, Mme Niamkhuu Ulambayar.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, si la loi Littoral du 3 janvier 1986, adoptée par le Parlement à l'unanimité, a fait l'objet de vifs débats par la suite, son bilan reste très positif. ans après son adoption, nous ne pouvons que constater ses bienfaits et son efficacité sur la protection des paysages et de la biodiversité. Elle a permis notamment de freiner la bétonisation des espaces proches du rivage et la dispersion des constructions dans les communes littorales. C'est la raison pour laquelle toute modification de ses équilibres doit être scrupuleusement pensée pensée en amont. a conduit le législateur à accorder progressivement des concessions, au fur et à mesure que l'on s'apercevait que le foncier de certains territoires se trouvait entièrement gelé, entravant ainsi toute possibilité de développement. Cela a justifié quelques entorses pour l'adapter aux réalités locales, notamment en ce qui concerne les installations de production d'énergies renouvelables, ces dernières nécessitant de la superficie. Nous avions évoqué le sujet dans cet hémicycle en janvier dernier, lors de l'examen de la proposition de résolution tendant au développement de l'agrivoltaïsme. À mon sens, les centrales au sol ne devraient être autorisées qu'exceptionnellement. Les panneaux photovoltaïques peuvent en effet être installés sur les toits des bâtiments ou en ombrières pilotables avec faible emprise au sol. Ces superficies, en particulier celles qui pourraient se situer en zone agricole, doivent être mises à l'abri de la convoitise d'éventuels promoteurs ou porteurs de projets peu soucieux de la vocation naturelle agricole des sols. Une position équilibrée, à la fois protectrice du littoral et des sols, ainsi que du droit pour tout territoire de participer à la transition énergétique doit être trouvée. Ce texte se limite à reprendre une disposition de la loi Climat et résilience censurée par le Conseil constitutionnel en vertu de l'article 45 de la Constitution. Que des panneaux photovoltaïques puissent être installés sur des sites dégradés ne soulève pas de difficultés. Je pense d'ailleurs que cette notion était préférable à celle de friches, celles-ci n'étant pas toujours dégradées. J'estime pour ma part que les terres agricoles ne devraient en aucun cas être considérées comme des friches, la priorité devant être d'accueillir les installations de production d'énergies renouvelables dans les zones artificialisées. Faut-il installer des centrales solaires à distance des agglomérations et des villages existants dans les communes littorales, comme le permettra la proposition de loi si elle est adoptée ? Rien n'est moins sûr, mais si cela peut accroître l'acceptabilité des projets photovoltaïques, soit Le recours à la procédure normale d'examen de la proposition de loi nous aurait permis d'avoir plus de recul. Dans le cadre de la procédure de législation en commission, nous sommes contraints d'accepter cette modification. Pourtant, rien ne servait de courir, alors qu'il est évident qu'à ce stade du calendrier parlementaire la proposition de loi ne sera pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avant la suspension des travaux. travaux. Nous nous contenterons donc des garde-fous qui ont été instaurés dès le départ et qui permettent de prévenir tout conflit d'usage : régime d'autorisation ; avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; obligation de réaliser une étude d'incidence prouvant que prouvant que la renaturalisation du site n'est pas plus pertinente que le projet proposé ; définition de la liste des friches envisagée après concertation avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. d'une nouvelle dérogation peut tout à fait s'entendre. Celle-ci apparaît cohérente dans la mesure où les éoliennes, dont l'impact paysager est plus important que les centrales photovoltaïques, et qui sont moins compatibles avec le voisinage des zones habitées, bénéficient d'ores et déjà d'une telle souplesse.

Néanmoins, si cette mesure permet à certaines collectivités locales, comme L'Île-d'Yeu, de s'inscrire dans un projet de renforcement de leur autosuffisance en matière énergétique, nous ne pouvons que soutenir cette démarche. Bien que ces dispositions, limitées à quelques zones identifiées, ne changent pas la donne quant à la diversification de notre mix énergétique, le groupe RDSE votera pour la présente proposition de loi. La parole

la loi Climat et résilience prévoyait le dispositif qui nous est aujourd'hui proposé, mais il a été censuré par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif. Passé à peu près inaperçu lors de l'examen du texte, cet ex-article 102 visait à permettre l'implantation de centrales solaires sur des friches situées en milieu littoral,

Sur le principe, nous partageons l'objectif de la proposition de loi, qui s'inscrit dans le principe de reconversion des friches, bien identifié par la commission d'enquête sur la pollution des sols, portée par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Parallèlement, nous souhaitons demeurer vigilants quant à la préservation des espaces littoraux. C'est la raison pour laquelle je me félicite de l'adoption de notre amendement visant à ce que le Conservatoire du littoral prenne une part décisive dans l'élaboration du décret listant les zones pouvant être concernées par un futur réaménagement photovoltaïque. Cette concertation obligatoire me paraît être un garde-fou bien plus efficace que l'étude d'incidence, qui, réalisée par le maître d'ouvrage, n'aura que très peu d'objectivité. En revanche,

il me semble que la droite sénatoriale et le Gouvernement commettent ici une erreur d'appréciation. Même si l'accord du maire, une autorisation d'urbanisme, reste nécessaire, il me semble qu'un vote des élus de la commune ou de l'EPCI concerné garantirait la transparence démocratique et favoriserait l'adhésion de la population au projet envisagé. Nous souffrons suffisamment de ce manque d'acceptabilité sociale des éoliennes pour risquer des réticences inutiles, faute de contrôle démocratique. À l'heure où la démocratie représentative pâtit d'une désaffection bien réelle, il m'apparaissait de bon droit d'impliquer en amont nos élus locaux dans ce type de décision, si importante pour notre avenir énergétique. Cette nouvelle exception- si j'ose dire -déroge enfin au parallélisme des formes, puisque l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme prévoit justement cette association des élus pour les éoliennes, celle-là même qui, dans le cas présent, fait défaut. Ne l'oublions pas, mes chers collègues, certains projets de centrale solaire seront bien acceptés, tandis que d'autres feront débat. C'est inévitable et je regrette que vous n'ayez pas entendu raison sur ce point. Nonobstant cette remarque de bon sens qui pourrait inspirer nos futurs députés, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera ce texte, car il adapte notre droit pour répondre à des attentes dans bon nombre de territoires, notamment insulaires, comme l'a souligné notre collègue Didier Mandelli. La jurisprudence administrative est constante sur ce sujet et interprète strictement la notion de continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Plusieurs autorisations de construire ont ainsi été annulées pour ce motif. Cette dérogation permettra donc d'éviter ce genre d'écueil auquel sont confrontés les élus et que j'ai bien connu à l'époque où à l'époque où j'étais maire des Ponts-de-Cé. J'ai en effet moi-même fait construire sur une ancienne décharge une centrale solaire, qui est la plus grande unité photovoltaïque de la région des Pays de la Loire : elle produit aujourd'hui 11 000 mégawatts par an, soit la consommation électrique de 4 000 foyers. ans, il aura fallu six ans pour obtenir les autorisations nécessaires de la CRE, alors que le site n'était même pas situé sur un littoral ! La France est en retard sur les énergies renouvelables et il s'agirait pour le Gouvernement de regarder en face

En conclusion, ce texte représente l'un des leviers utiles que nous pouvons actionner pour intensifier la production électrique d'origine solaire dont notre pays a besoin. Ne boudons pas notre unanimisme pour adopter cette proposition de loi, même si, je le répète, la voix de la démocratie représentative doit figurer dans cette nouvelle dérogation à la loi Littoral pour emmener le plus grand nombre dans la transition écologique. La parole

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art, présentée il y a deux ans, connaît aujourd'hui son aboutissement, après un long, mais fructueux travail parlementaire, qui a permis de l'enrichir considérablement. Je m'en réjouis. Il faut rendre hommage à celles et à ceux dont la détermination a permis l'émergence de points de consensus par-delà les clivages politiques.

et Belrhiti, ainsi que tous les sénateurs et députés qui ont permis à ce texte de connaître une issue favorable. Parmi eux, je pense tout particulièrement au député Maillard, dont le travail a été décisif. Ce texte est, en effet, le fruit d'un minutieux travail de concertation et de coconstruction mené avec les professionnels du secteur et le Conseil des ventes volontaires. Je tiens là aussi à saluer l'implication et le sens du dialogue de toutes les parties intéressées, sans lesquelles ce travail n'aurait jamais pu aboutir. Cette réforme dessine des lignes de force pour l'avenir de la profession d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Elle répond aux préoccupations exprimées dans l'excellent rapport réalisé par Mme Henriette Chaubon et M. Édouard de Lamaze, dont les réflexions ont apporté un éclairage précieux et que je souhaite également remercier chaleureusement. Cette réforme permettra aux opérateurs de ventes volontaires de retrouver une dénomination qui leur est familière et qui est en réalité la dénomination historique de leur profession : celle de commissaires-priseurs, exerçant au sein de maisons de vente. Cette réforme rénove également en profondeur la gouvernance de la profession. Elle remplace le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par une nouvelle autorité de régulation dont les compétences sont élargies : le Conseil des maisons de vente. La composition de cette instance a fait l'objet de discussions nourries et indubitablement utiles. Je crois qu'un bon équilibre a été trouvé : les membres de la profession y seront majoritaires d'un siège- six membres sur mais le président de la formation sera nommé par le garde des sceaux parmi les personnalités qualifiées. Les prérogatives du futur Conseil des maisons de vente seront également renforcées. Il est en effet important que ce Conseil demeure un organe régulateur de la profession, et non un syndicat ou un ordre professionnel. La réforme refonde aussi le régime disciplinaire applicable aux professionnels du secteur. C'est un point important. Un régime disciplinaire efficace est en effet un gage de crédibilité pour le marché des ventes volontaires. Vous savez que la modernisation du régime disciplinaire des professions est une question qui m'est chère. La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a procédé à la modernisation de la déontologie et de la discipline des professions du droit, qu'il s'agisse des avocats ou des officiers ministériels. Je me réjouis de voir la profession des opérateurs de ventes volontaires prendre le même chemin. La profession d'opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sortira renforcée de cette réforme, qui lui ouvre de nouveaux domaines d'intervention, comme les inventaires fiscaux, la vente de biens incorporels ou encore les ventes des biens des mineurs sous tutelle. Le marché des ventes volontaires est une composante essentielle du marché de l'art français. Il faut soutenir son développement et nourrir l'ambition qu'il demeure un facteur d'attractivité pour notre pays. Enfin, je me réjouis que le travail de concertation conduit à l'occasion de l'élaboration de la proposition de loi ait permis de régler la question de la poursuite d'activité, après le 1 juillet 2022, de la quarantaine d'huissiers de justice qui, depuis plusieurs années, réalisent de façon régulière des ventes volontaires dans leur office. L'ensemble des améliorations apportées au texte a fait l'objet- je le sais -de discussions approfondies entre les deux assemblées, afin de parvenir à un compromis de nature à permettre l'adoption définitive de la proposition de loi cet après-midi. je ne peux à cet égard que saluer le travail accompli, notamment celui de votre commission des lois, qui a adopté le texte de l'Assemblée nationale sans modification, mais après des échanges nourris avec les députés.

Le Gouvernement ne peut que se féliciter que, sur un sujet aussi important que la défense et la modernisation du marché de l'art français, le travail conjoint des deux assemblées ait pu aboutir à ce beau résultat, au terme de l'actuelle mandature.

plus de deux ans après sa première lecture par le Sénat, la proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art, dont notre collègue Catherine Morin-Desailly est à l'origine, arrive au terme de son examen parlementaire. La commission des lois se félicite de voir aboutir cette initiative sénatoriale particulièrement bienvenue. Grâce à ce texte, un vent nouveau de liberté viendra souffler sur un secteur d'activité dont le poids dans l'économie française n'est pas négligeable et qui participe également au rayonnement culturel de notre pays. Cette proposition de loi a pour objet de réformer le système de régulation et, plus largement, le régime légal des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dont la vente d'objets d'art et de collection représente environ la moitié. Alors que Paris était, dans les années 1950, la capitale mondiale des ventes aux enchères, notre pays n'occupe plus aujourd'hui que le quatrième rang international, loin derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et, désormais, la Chine. Chine. Ce recul n'est pas inéluctable, toutefois, à condition que nous sachions accompagner le renouvellement de la profession. Les ventes volontaires de meubles aux enchères ont été progressivement libéralisées, depuis le début des années 2000, sous l'effet du droit européen. Elles constituent néanmoins toujours une profession réglementée. Or la législation en la matière reste inutilement restrictive et freine la modernisation du secteur. Initialement, la proposition de loi de Catherine Morin-Desailly avait pour objet exclusif de réformer l'autorité de régulation de ce secteur d'activité. Malgré les qualités personnelles de ses membres et de ses présidents successifs, le Conseil des ventes volontaires n'a pas donné entière satisfaction. Sa gestion a longtemps été jugée dispendieuse, ce qui lui a attiré les critiques de la Cour des comptes. Surtout, les professionnels reprochent au Conseil des ventes volontaires, non sans quelque apparence de raison, d'exercer un contrôle inutilement tatillon de leurs activités, sans parvenir à empêcher les quelques scandales qui défraient occasionnellement la chronique. L'une des compétences les plus importantes du Conseil vient d'ailleurs de lui être retirée, parce qu'il ne l'exerçait pas convenablement : je veux parler du contrôle du respect, par les opérateurs, de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, compétence qui a été transférée à la direction générale des douanes et à la Commission nationale des sanctions. À dire vrai, l'on pourrait s'interroger sur la nécessité de maintenir une autorité de régulation propre au secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères. Une telle autorité n'existe dans aucun autre pays d'Europe. En France même, il n'en existe pas dans des secteurs d'activité connexes, par exemple le commerce d'oeuvres d'art. Bien sûr, des contrôles sont nécessaires, notamment pour prévenir les risques spécifiques de fraude liés au procédé des enchères.

qui ne fait pas consensus. Elle a, en revanche, approuvé le choix de réformer en profondeur l'autorité de régulation existante. La proposition de loi prévoit d'instituer, en lieu et place du Conseil des ventes volontaires, un Conseil des maisons de vente, qui conserverait le caractère d'une autorité de régulation, mais qui verrait ses missions élargies à la promotion des ventes aux enchères, à l'information sur la réglementation applicable et au règlement amiable des différends. La composition de cette instance serait profondément modifiée. Son collège serait désormais constitué en majorité de représentants élus par les professionnels du secteur, de manière à assurer une représentation équilibrée du territoire français. En première lecture, le Sénat a prévu que le président du Conseil des maisons de vente soit nommé parmi les membres du collège et sur proposition de celui-ci. Dans un souci d'équilibre, les députés ont estimé préférable que le président soit choisi parmi les membres nommés et ont donc supprimé le pouvoir de proposition du collège. La commission des lois n'a pas remis ce choix en question. La proposition de loi prévoit aussi de rénover les conditions d'exercice, par le Conseil des maisons de vente, Le pouvoir disciplinaire serait désormais exercé par une commission des sanctions, distincte du collège, et le régime des sanctions serait modifié, notamment avec l'introduction d'une sanction pécuniaire. Sur ce point, je me félicite que les députés, après avoir envisagé de transférer les attributions disciplinaires du Conseil au tribunal judiciaire de Paris, aient finalement rétabli un texte très proche de celui qu'a adopté le Sénat en première lecture. Au-delà de cette réforme de l'autorité de régulation, la proposition de loi a été notablement enrichie, en première lecture, grâce au travail de notre ancienne collègue Jacky Deromedi, qui était alors rapporteur de la commission de lois. Je veux ici lui rendre hommage. Sans entrer dans le détail, je mentionne toutefois quelques-uns de ces ajouts. L'un d'entre eux, qui peut paraître technique, revêt pourtant une importance considérable : il s'agit de l'article 3, qui étend aux meubles incorporels le régime légal des ventes volontaires de meubles aux enchères. Cette innovation tombe à point nommé pour accompagner le développement fulgurant du marché des oeuvres d'art numériques, notamment des NFT (), ces « jetons » représentatifs de fichiers numériques individualisés. Une oeuvre entièrement numérique de l'artiste américain Beeple, consistant en un assemblage de 5 000 dessins, a par exemple été vendue 69 millions de dollars l'an dernier chez Christie's à New York, sous forme de NFT. Une telle vente n'aurait pas été possible en France, en raison de la législation applicable. Plus largement, grâce à cet apport majeur du Sénat, les maisons de vente françaises verront s'ouvrir à elles de nouveaux marchés, appelés à se développer avec l'essor de l'économie de l'immatériel vente aux enchères de dessins et de modèles, de brevets, de marques, mais aussi de fonds de commerce ou de clientèles civiles, etc. Plusieurs autres articles ont également pour objet d'étendre le champ d'activité potentiel des opérateurs de ventes volontaires en leur permettant de procéder aux inventaires fiscaux en cas de succession, grâce à une initiative de Jean-Pierre Sueur, mais aussi en les habilitant à réaliser certaines catégories de ventes aujourd'hui classées parmi les ventes judiciaires. D'autres dispositions visent à réduire les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur nos maisons de vente, en allégeant le formalisme auxquelles elles sont soumises, lorsqu'elles réalisent des ventes de gré à gré, ou encore en leur permettant de regrouper leur livre de police et leur répertoire des procès-verbaux. Enfin, nous avions souhaité garantir une concurrence équitable dans le secteur des ventes de meubles aux enchères, en soumettant les notaires qui souhaitent réaliser de telles ventes, comme ce sera bientôt le cas pour les commissaires de justice, à l'obligation de constituer à cet effet une société distincte de leur office et à une obligation de qualification renforcée. L'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions, ce que je m'explique assez mal. Il faudra y revenir, monsieur le garde des sceaux, car l'Autorité de la concurrence nous a alertés sur cette inégalité injustifiée. Dans l'ensemble, le texte adopté par les députés ne remet pas en cause les orientations de la réforme voulue par le Sénat. C'est pourquoi, mes chers collègues, la commission des lois vous propose de l'adopter sans modification, afin qu'il puisse entrer en vigueur sans plus tarder. je tiens à rassurer mes collègues alsaciens-mosellans : cette proposition de loi n'aura aucune incidence sur le droit local. En Alsace-Moselle, les ventes volontaires de meubles aux enchères sont régies par le droit commun. C'est au sujet des ventes judiciaires que le droit local s'écarte du droit commun, puisqu'il n'existe pas de commissaires-priseurs judiciaires en Alsace-Moselle. Les notaires et les huissiers de justice en font office. La parole est à M.

nous sommes réunis cet après-midi afin d'examiner la proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art, plus de deux ans après son adoption en première lecture par la Haute Assemblée. Dans le paysage mondial des ventes aux enchères, la France occupe une place particulière depuis le XVI siècle. Toutefois, si, jusqu'à la fin des années 1950, elle a été première en concentrant 60 % du marché mondial d'oeuvres d'art, elle n'en représente actuellement plus que 6 % et se situe au quatrième rang mondial, loin derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. Le secteur des ventes volontaires aux enchères publiques a été peu à peu libéralisé au début des années 2000, avec la fin du monopole des commissaires-priseurs, la suppression de leurs offices ministériels, le passage à un régime d'agrément, puis à un simple régime de déclaration préalable des opérateurs.

Malgré cela, le retard du marché français persiste : un certain nombre d'insatisfactions et d'inquiétudes ont été exprimées, notamment sur la fin du monopole des commissaires-priseurs ou sur la soumission au contrôle d'un organe de régulation extérieur à la profession. C'est pourquoi cette proposition de loi a pour objectif de redynamiser l'ensemble du secteur des ventes volontaires en France. Initialement, ce texte ne comportait qu'un article unique visant à réformer en profondeur le système français de régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères, en modifiant la dénomination, la composition, les missions et le fonctionnement de l'actuel Conseil des ventes volontaires. L'instauration d'un Conseil des maisons de vente composé majoritairement de représentants élus de la profession donne un rôle prépondérant à cette autorité modernisée, au service non seulement des professionnels des ventes volontaires, mais également des vendeurs et des acheteurs, qui font vivre le marché de l'art. Je tiens à souligner que le Sénat a enrichi la proposition de loi en première lecture et qu'au cours de la navette les deux assemblées ont trouvé des points de convergence. Aussi, j'approuve la position de notre commission des lois, qui n'a pas souhaité déposer de nouveaux amendements, afin de parvenir à un vote conforme. J'espère que cet esprit consensuel prévaudra à l'issue de l'examen de Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, cette proposition de loi concrétise un objectif de modernisation et de régulation du marché de l'art. Elle permettra de redonner un nouveau souffle aux maisons de vente et à la profession de commissaire-priseur. Elle contribuera à mieux les armer face à la compétition internationale. Aussi, le groupe Les Indépendants -République et Territoires votera en faveur de ce texte très attendu par l'ensemble des acteurs du secteur des ventes volontaires.

cela a été dit, la place française a perdu au fil du temps sa position face aux États-Unis et à la Chine, au point de faire de la France un acteur minoritaire du marché de l'art mondial alors qu'elle a occupé la première place dans les années 1950. Même si la France reste leader dans certains domaines comme le design, les manuscrits et les arts premiers, elle est devenue un acteur secondaire sur les marchés les plus porteurs comme l'art contemporain, l'art moderne et l'impressionnisme. Notons toutefois que le produit des ventes aux enchères publiques en France a atteint en 2021, selon les premiers chiffres publiés par le Conseil des ventes, le montant record de 4 milliards d'euros, soit une augmentation de près de 40 %. Dans ce contexte, la France devrait confirmer sa quatrième place sur le marché mondial. Les maisons de ventes aux enchères en France connaissent donc une sortie de crise spectaculaire, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter collectivement. Cette dynamique doit nous inciter à poursuivre notre travail pour donner un souffle nouveau à cette profession, offrir aux maisons de ventes volontaires de nouveaux champs d'activité possibles et les encourager à consolider leurs structures. Il convient toutefois de préserver ce qui constitue les conditions de l'excellence française, reconnue de tous, lesquelles expliquent la confiance dont jouissent ces professions de la part des clients étrangers : l'autorité de régulation- le Conseil des ventes volontaires -, qui garantit la sécurité des ventes et prémunit

Les représentants des professionnels occuperont donc la majorité des sièges, soit six des onze sièges. Cette composition pose la question de l'assimilation du Conseil à un ordre professionnel, en raison de la présence majoritaire de professionnels au sein de la structure, d'une part, de leur élection par leurs pairs,

des informations transmises au Conseil. Le maintien d'un véritable régulateur du marché, tiers de confiance indépendant veillant à la transparence du processus d'enchères et à la protection des acheteurs et des vendeurs, commande que ce Conseil reste majoritairement composé de non-professionnels ou, au moins, que ces derniers soient à égalité de sièges. Or, l'existence du régulateur est l'un des fondements de la réglementation. Craignant de mettre en place un nouvel ordre professionnel pouvant contrevenir au droit communautaire, vous avez créé un nouvel organe distinct, dénommé « commission des sanctions », qui exercera ce pouvoir disciplinaire. Espérons

une maison des ventes volontaires et ont déjà exercé ce métier. Ainsi, ceux qui, de 2016 à 2021, ont tenu au moins vingt-quatre ventes sur au moins trois années consécutives ou effectué des vacations d'un montant total de 230 000 euros seront dispensés non seulement de formation, mais aussi d'examen. Rappelons ici que cette disposition leur avait été refusée par le Conseil d'État. Il est fort à craindre que cette disposition ne crée dans nos territoires une situation extrêmement concurrentielle, laquelle ne sera pas sans conséquence. Mes chers collègues, nous partageons le même objectif. Il s'agit de préserver l'attractivité économique de la profession et de réfléchir à son adaptation

le présent texte porte sur l'amélioration du système de régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, soit principalement des oeuvres d'art, mais aussi toutes sortes d'objets mobiliers, y compris des machines industrielles et même des animaux, notamment des chevaux, comme l'a rappelé notre rapporteure. Notre assemblée avait dès 2018 travaillé sur l'attractivité et la compétitivité juridique du marché de l'art français. En quelques décennies, le marché de l'art est devenu très concurrentiel. Les opérateurs français des ventes volontaires ont ainsi dû s'adapter à un phénomène d'internationalisation qui a précipité le déclin de l'attractivité de la France, longtemps réticente aux évolutions. En parallèle d'un contexte concurrentiel international accru, les maisons de ventes doivent faire face à l'émergence du e-commerce et de sites d'annonces commerciales en ligne. Dans les années 1960, notre pays représentait encore 60 % du marché mondial de l'art ; il n'en représente plus que 6 % aujourd'hui. Les raisons en sont multiples. Elles sont d'ordre artistique, fiscal et administratif. Lors des auditions de la commission, plusieurs pistes ont été proposées, notamment l'évolution du Conseil des ventes volontaires,

Le grand mérite de ce texte est bien de renforcer la présence des professionnels du marché de l'art au sein de ce Conseil afin que ce dernier puisse faire le lien entre les artistes et les autorités de régulation, à l'image du ministère de la culture.

De plus, au vu du faible nombre de contentieux, et afin de prévenir au mieux l'apparition de conflits d'intérêts, il semble cohérent de remettre ce pouvoir au tribunal judiciaire de Paris et de ne pas faire de ce Conseil une instance ordinale. Son rôle doit être d'édicter et de promouvoir de bonnes pratiques et des obligations déontologiques. saluons également le transfert des missions de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à la direction générale des douanes et droits indirects. Enfin, ce texte permet une remise à plat et une grande simplification de l'environnement du marché de l'art. Nous saluons à la fois la simplification des démarches, notamment la suppression de l'établissement d'un mandat de vente par écrit et d'un procès-verbal de la cession et le rétablissement d'une concurrence équitable entre notaires et autres vendeurs, et la volonté d'instaurer une formation continue pour les commissaires-priseurs. Reste toujours la problématique des ventes non régulées en ligne et de la double exigence de protection des usagers, des acheteurs comme des vendeurs, et surtout de compétitivité du secteur. La transformation numérique du secteur et son encadrement demeurent un enjeu.

Un marché de l'art ne peut vivre qu'avec un vivier bouillonnant de talents. Le secteur de la culture a été très affecté par la crise sanitaire. Le plan de relance n'est pas à la hauteur des enjeux dans une nation de culture ouverte à tous les artistes. Il ne permettra pas à ces derniers de s'affranchir des règles du marché.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la loi du 10 juillet 2000 a abrogé le monopole des commissaires-priseurs et a institué les sociétés de ventes volontaires,

Le commissaire-priseur est de moins en moins un officier ministériel chargé par l'État d'une mission de service public. Il convient donc de se demander si ces ventes volontaires doivent néanmoins continuer d'être encadrées par la puissance publique. Autrement dit, la fin d'une profession réglementée impose-t-elle la libéralisation du secteur économique qu'elle animait ? Il faut reconnaître que, depuis la loi du 10 juillet 2000, le marché de l'art s'est profondément transformé, dans un sens qui était prévisible. Trois grandes maisons de ventes s'approprient aujourd'hui plus de la moitié du volume des ventes et les anciennes maisons françaises ont toujours plus de difficultés à résister à cette concentration qui peut demain les emporter. La présente proposition de loi déposée par notre collègue Catherine Morin-Desailly s'inspire des rapports et des évaluations suscités par ces évolutions très rapides et se justifie par la perte d'influence de la place de Paris. Elle s'attache principalement à corriger le mode de fonctionnement et les attributions du Conseil des ventes volontaires. Ces mesures techniques vont dans le bon sens et renforcent quelque peu l'encadrement de cette activité. Néanmoins, notre collègue Catherine Catherine Morin-Desailly souhaite que ce Conseil des ventes volontaires rénové soit « au service d'une profession portant un niveau élevé d'exigence de probité et d'expertise ». Je partage totalement son ambition. J'entends parfois exprimer l'idée selon laquelle l'attractivité du marché parisien pourrait être mieux défendue si ce dernier bénéficiait de la même déréglementation que ses concurrents à l'étranger. Je suis intimement convaincu du contraire et je pense que les garanties supérieures qu'il peut offrir à ses clients lui profiteront nécessairement un jour. Nous venons de voter la restitution d'un tableau de Maurice Utrillo aux ayants droit de Georges Bernheim. Achetée à une grande maison de vente londonienne par la ville de Sannois, cette oeuvre avait été spoliée par l'organisation nazie Rosenberg. Le vendeur refuse toute indemnisation, estimant qu'il ne pouvait disposer d'information sur ce vol. Ainsi que l'a justement dénoncé, à cette même tribune, mon collègue Sébastien Meurant, il n'est pas acceptable qu'une maison internationale aussi prestigieuse dégage sa responsabilité de la sorte. L'an passé, le bureau parisien de la plus grande société de vente aux enchères, dont le siège est à Londres, a dispersé soixante oeuvres d'Afrique et d'Océanie de la collection de Michel Périnet, pour 66 millions d'euros. Les conditions de l'acquisition de toutes ces pièces n'ont pas été établies avec précision. Alors qu'il est demandé aux musées nationaux de restituer les oeuvres acquises par la violence et de réaliser un travail de récolement des provenances, comment peut-on admettre que des maisons de vente s'affranchissent de ces vérifications indispensables ? Après cette révision modeste de la loi de 2011, il faut engager une réflexion plus globale sur le marché de l'art. À tout le moins, la France doit ratifier sans délai la convention

je suis très heureuse que le Sénat examine aujourd'hui en deuxième lecture ma proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art. Voilà bientôt quatre ans, en mars 2018, que notre chambre s'est saisie de ce sujet, inquiète de la perte de compétitivité de la France dans ce secteur. En tant que présidente de la commission de la culture, j'avais alors organisé avec mon collègue Philippe Bas, président de la commission des lois, deux tables rondes consacrées à l'attractivité du marché de l'art avec des représentants des professionnels et des instances de régulation et de contrôle. Nous avions pu alors repérer un certain nombre de blocages, certains d'ordre fiscal et réglementaire, mais aussi plusieurs rigidités administratives susceptibles de corseter le développement du marché de l'art en France. Le constat était aussi que la libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques engagée par les réformes de 2000 et de 2011 pour se mettre en conformité avec le droit européen n'avait pas eu sur le terrain les effets escomptés, malgré la progression sensible du volume des ventes aux enchères réalisées depuis lors. Plusieurs études faisaient état des difficultés rencontrées par les professionnels en raison de l'arrivée d'autres acteurs sur le marché, d'une concurrence internationale croissante, mais aussi des conséquences de la réforme des commissaires de justice. Dès lors, il fallait poursuivre la réforme, l'enjeu étant de concilier une plus grande liberté sur le marché des ventes volontaires avec le nécessaire maintien d'une régulation, gage de crédibilité et de probité dans un secteur imposant une grande attention et une véritable rigueur au regard des risques de fraudes qui peuvent le traverser. La réforme du Conseil des ventes alors proposée, soutenue par de très nombreux collègues, a bénéficié des échanges nourris que j'ai pu avoir avec Henriette Chaubon et Édouard de Lamaze, auteurs de l'excellent rapport commandé par la suite par l'ancienne garde des sceaux, elle-même alertée des difficultés de la profession. Cette réforme est substantielle, car elle modifie la composition, l'organisation interne, les missions et jusqu'à la dénomination du Conseil pour en faciliter l'identification. D'aucuns s'interrogent sur le mélange des professionnels et des magistrats. à noter que toutes les réformes des professions régulées depuis dix ans ont été réalisées sur le mode de l'échevinage, reposant sur de nouveaux équilibres entre le caractère professionnel et la fonction de régulation. Sitôt voté en octobre 2019, enrichi de plusieurs autres dispositions par notre commission des lois pour accroître et simplifier l'activité des opérateurs de ventes, ce texte a été transmis à l'Assemblée nationale. Malheureusement, son examen a été stoppé par la crise sanitaire au début de l'année 2020. Depuis lors, avec mon collègue Sylvain Maillard, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, avec qui nous avons travaillé en bonne intelligence, nous n'avons eu de cesse de solliciter du Gouvernement sa réinscription à l'ordre du jour. Nous y sommes enfin ! C'est un élément de satisfaction, d'autant que les députés ont validé l'essentiel du texte transmis par le Sénat. Les modifications essentiellement techniques et rédactionnelles apportées ont fait l'objet d'échanges avec l'Assemblée nationale et la Chancellerie pour aboutir à une écriture satisfaisante pour tous. Seul changement majeur : le mode de désignation du président du nouveau Conseil, dont nous avions beaucoup débattu ici en première lecture, sachant que la navette nous donnerait l'occasion d'approfondir la réflexion et de parvenir à un équilibre. L'essentiel du texte issu du Sénat reste sinon inchangé. la nouvelle composition du Conseil permettant une présence accrue des professionnels tout en assurant la représentation du maillage territorial et des autorités de régulation ; l'élargissement du périmètre des missions du Conseil pour en faire un véritable outil de concertation entre le Gouvernement et les professionnels la fonction disciplinaire du Conseil. Pour ma part, j'étais très attachée à la création d'un organe disciplinaire indépendant au sein du Conseil, estimant qu'il serait contre-productif, compte tenu du fort encombrement de la justice, de renvoyer cette fonction vers les tribunaux. Cette option permet par ailleurs le recours à la médiation. Cette réforme très attendue permet donc la création d'un Conseil au service d'une profession portant un niveau élevé d'exigence de probité et d'expertise, comme l'a relevé Pierre Ouzoulias. À cet égard, on notera que, grâce au Sénat, les personnes physiques habilitées à diriger des ventes volontaires vont retrouver le beau titre de « commissaire-priseur », aussitôt que la profession de commissaire-priseur judiciaire aura disparu pour être fusionnée avec celle d'huissier de justice.

concentration du marché. Cette proposition de loi n'a aucune prétention à relancer à elle seule la compétitivité de la France sur le marché de l'art, ce serait très présomptueux. Il y aurait bien d'autres mesures à prendre. Je déplore, comme vous, mes chers collègues, que la France, si longtemps patrie de la création artistique, ne puisse plus dans le domaine de l'art bénéficier de la même activité qu'autrefois, mais notre pays dispose encore d'atouts considérables sur ce marché : la richesse formidable et inégalée de son patrimoine, les compétences et la formation des professionnels, ainsi que l'ancrage territorial des sociétés de ventes volontaires. Alors, restons

Je m'étonne et je me préoccupe en effet de l'opposition à ce texte de l'actuel président du Conseil des ventes, qui a pourtant été nommé par votre prédécesseur pour mettre en oeuvre la réforme. Il est pour le moins déplacé qu'il prenne aujourd'hui à partie les membres du CVV, qu'il leur adresse ses critiques et qu'il ait inscrit un vote sur le texte à l'ordre du jour de l'assemblée du CVV de jeudi dernier, vote qu'il a finalement et heureusement retiré. Et encore, je n'ai pas tout dit Jusqu'à preuve du contraire, mes chers collègues, les décisions appartiennent toujours au Gouvernement et au Parlement souverain dans la fabrique de la loi. Faut-il en plus rappeler, comme vous l'avez fait, monsieur le garde des sceaux, que ce texte a été voté à l'unanimité par les deux chambres ? C'est suffisamment rare pour être souligné. Nous resterons donc très vigilants. Nous savons

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la France, considérée hier comme la principale place du marché mondial de l'art, serait aujourd'hui déclassée. On ne peut le nier, notre pays n'est plus le leader qu'il était dans les années 1950, quand ses acteurs dominaient encore 60 % du marché. Néanmoins, selon les classements, il se maintient à la quatrième ou sixième place. Dans un monde de plus en plus ouvert, ce peut être le signe d'une vitalité à soutenir. Doit-on juger la valeur d'une place à l'aune des transactions les plus folles qui se croisent entre New York, Londres et Pékin ? En 2019, le, un lapin d'acier de Jeff Koons, vendu à plus de 91 millions de dollars, n'a sans doute pas manqué à lui seul de doper le marché américain La même année, la France vendait presque autant de lots que l'Oncle Sam. Le volume est un indice tout aussi important que la valeur, d'autant que la formation des prix de l'art conserve sa part de mystère. Et je ne parlerai pas des scandales qui entachent régulièrement certaines grosses transactions La France conserve ses atouts majeurs : une longue histoire, un patrimoine riche et solide et une politique muséale, qui participent de l'attractivité du marché de l'art. Chaque facette est complémentaire de l'autre, au point que les commissaires-priseurs se définissent bien souvent comme des passeurs de l'histoire. J'en viens ainsi à la proposition de loi, qui concerne en particulier le secteur des ventes volontaires aux enchères publiques, dont les commissaires-priseurs sont les premiers acteurs. En première lecture, le groupe RDSE avait approuvé le texte déposé par notre collègue Catherine Morin-Desailly, qui vise principalement à modifier le système de régulation de ces ventes. À ce stade, il apparaît qu'un équilibre a été trouvé avec nos collègues députés pour redonner du souffle au Conseil des maisons de vente. Une majorité de professionnels en son sein, plus de diversité territoriale, un pouvoir disciplinaire exercé par un organe distinct, la commission des sanctions : toutes ces dispositions vont dans le bon sens. La commission des lois semble se satisfaire de l'évolution de la proposition de loi, qui par ailleurs prend acte du nouveau statut de commissaire de justice. Mon groupe se range à son avis. avis. Nous comprenons bien aussi que ce texte ne représente qu'un seul volet des politiques de soutien au marché de l'art. Aujourd'hui, j'en évoquerai un autre : la fiscalité liée aux oeuvres d'art. Mettre en place une fiscalité attractive pour encourager la circulation et l'acquisition des oeuvres est un outil intéressant, à deux conditions. La première est de mesurer régulièrement l'effet concret des dispositifs fiscaux qui profitent tant aux entreprises qu'aux particuliers. seconde, essentielle, est de vérifier que la fiscalité applicable aux oeuvres d'art ne constitue pas seulement un effet d'aubaine pour certains contribuables et que les conditions de son recouvrement ne conduisent pas à des évaluations discutables. Monsieur le garde des sceaux, ce volet mérite réflexion. Par ailleurs, il a manqué dans la discussion de ce texte un plus grand débat sur le rôle qu'auront à jouer dans le futur de l'art les NFT. Ces jetons non fongibles sont les certificats de propriété d'une oeuvre numérique. Alors que nous allons par cette proposition de loi en faciliter les enchères, nous devons nous interroger sur l'apport à l'humanité des produits de la et de l'économie immatérielle. À l'heure où la France et le monde doivent redoubler d'efforts pour sauver la planète, cette économie du vide doit nous alerter. Conscients des limites planétaires, allons-nous créer de la richesse pour créer de la richesse, sans nous interroger sur les effets sur l'environnement de nos actions ? prêté la Joconde aux Américains en 1963, le président Pompidou a rappelé que la possession de chefs-d'oeuvre imposait de grands devoirs. L'amélioration des outils du marché de ventes aux enchères en fait partie, les maisons de vente constituant une belle vitrine pour le rayonnement culturel de la France dans le monde.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l'art et l'argent : vaste sujet ! Ah ! On pourrait même dire, madame le rapporteur : l'art, l'argent, le pouvoir Combien de peuples, de cultures, de civilisations ont été spoliés au fil du temps ? Combien d'oeuvres

il y a là matière à une vaste réflexion. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet, comme il l'a lui-même suggéré. En attendant, chère Catherine Morin-Desailly, vous nous avez présenté un texte dont vous avez eu la lucidité de nous dire qu'il ne constituait pas une révolution. D'ailleurs, il faut toujours préférer les réformistes qui font des réformes aux révolutionnaires qui ne font pas la révolution ! Bravo ! M. le garde des sceaux approuve l'en remercie ! Ce texte, en cette époque où le marché de l'art ne représente en France que 6 % du marché mondial, comporte plusieurs avancées qui seront utiles. Je pense tout d'abord à la transformation du Conseil des ventes volontaires en un Conseil des maisons de vente,

les professionnels représentant leurs collègues au sein de ce Conseil, nous avions pensé que son président aurait pu être nommé en son sein par le Gouvernement, mais l'Assemblée nationale a été d'un autre avis. Elle a préféré que le président soit choisi parmi les membres nommés

des pouvoirs publics. Nous pourrions en discuter longtemps. Toujours est-il qu'il est apparu préférable à notre commission, et je pense qu'elle a eu raison, de proposer l'adoption conforme de ce texte plutôt que de le renvoyer à une prochaine lecture, qui, sans doute, n'aurait jamais eu lieu, ce qui eût été très dommageable.

capitale. L'allégement des formalités des ventes de gré à gré ou l'accès partiel des ressortissants européens à certaines ventes sont,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier le président Retailleau et le groupe Les Républicains d'avoir inscrit à notre ordre du jour ce débat sur le bilan des politiques éducatives du quinquennat. Fait rare, vous êtes, monsieur le ministre, le seul titulaire depuis cinq ans du portefeuille de l'éducation nationale. Et ces cinq années vous ont permis d'engager de nombreuses réformes : scolarité obligatoire dès trois ans, priorité au primaire, refonte du baccalauréat, revalorisation du métier de professeur, réorganisation systémique de l'école inclusive. fait preuve d'une vraie volonté réformatrice. Mais celle-ci a-t-elle eu sur l'école l'effet de revitalisation escompté ? En fait, à l'heure du bilan, une seule question vaut : l'école se porte-t-elle mieux aujourd'hui qu'il y a cinq ans ? Tentons de le mesurer au travers de quatre orientations : la transmission des savoirs fondamentaux, la fluidité des parcours entre les enseignements scolaire et supérieur, le regard de la société sur les professeurs et l'autonomie des établissements. Nous donnerons la priorité à l'école primaire, pour que tous les élèves sachent lire, écrire et compter en arrivant en sixième. » Pourtant, en septembre dernier, 28 % des élèves de sixième ne disposaient toujours pas d'une compréhension suffisante en mathématiques.

», et il n'a « aucun effet supplémentaire en cours élémentaire, où le différentiel de progression est, en français comme en mathématiques, faible et non significatif ». Les écarts entre les élèves relevant de l'éducation prioritaire et les autres continuent donc de se creuser. L'école de notre pays n'a pas inversé une tendance lourde à une transmission de plus en plus aléatoire des savoirs fondamentaux, en particulier pour les élèves des quartiers les plus défavorisés. La fluidité des parcours entre l'enseignement scolaire et supérieur constituait une autre de vos ambitions en 2017. La réforme du baccalauréat devait y pourvoir. La liberté de choix accordée aux lycéens est certes intéressante, mais les modalités d'organisation restent compliquées. Professeurs et parents regrettent une course permanente à l'évaluation. Le très grand nombre de spécialités et d'options augmente les inégalités entre les petits et les grands lycées. Surtout, les élèves peu ou mal conseillés s'aventurent parfois dans des appariements de spécialités sans cohérence avec les attendus et les prérequis de l'enseignement supérieur. Celui-ci ne s'est d'ailleurs que très partiellement adapté à la réforme du baccalauréat, créant bien des angoisses chez les lycéens- et c'est une attitude qui n'est pas acceptable. Une meilleure articulation entre lycée et licence se dessine-t-elle ? On peut en douter. Enfin, le baccalauréat à la carte a mis en difficulté l'enseignement des mathématiques : 31 % des lycéens de première et de terminale générales ne suivent plus aucun enseignement dans cette discipline, avec des contrastes entre garçons et filles indignes de notre pays. Moins performante dans la transmission des savoirs fondamentaux, et n'ayant guère amélioré la fluidité des parcours entre le scolaire et le supérieur, l'école est également moins considérée, moins respectée. Un sondage commandé par le Sénat à l'occasion de l'Agora de l'éducation le montre nettement : 53 % des Français estiment que l'école fonctionne mal, et 65 % sont pessimistes sur son avenir, une proportion qui atteint presque 80 % chez les enseignants. Sur ce point, toutes les études démontrent que vous n'avez pas réussi à mener l'immense chantier qui s'offrait à vous. Désormais, dans le pays où Victor Hugo assimilait les maîtres d'école à « des jardiniers en intelligence humaine », seuls 7 % des professeurs de collège estiment que leur profession est appréciée. Vous vouliez pourtant redonner toute sa place au professeur dans sa classe et dans la société. Or la revalorisation salariale s'est enlisée dans un saupoudrage empêchant de reconnaître ceux qui s'engagent au-delà de leurs strictes obligations. Quelque 1 500 d'entre eux sont Les jeunes aspirants enseignants rechignent de plus en plus à se retrouver dans les établissements et les quartiers les plus difficiles, alors que la progression de la violence à l'école n'a pas été enrayée et que des établissements de plus en plus nombreux sont chaque jour davantage soumis aux pressions communautaires. À ces difficultés s'ajoute enfin un pilotage dont la verticalité est contestée par les syndicats et les personnels. N'aviez-vous pas annoncé, en 2017, vouloir donner « plus d'autonomie aux équipes éducatives » fait, seulement 2 % des décisions prises dans les établissements le sont en autonomie totale, comme vient de le signaler un rapport de la Cour des comptes. Ce quinquennat n'aura donc été en rien celui d'une rupture avec une pratique très jacobine du pilotage. Bien au contraire, il n'y a jamais eu autant de discours prescriptifs, de circulaires, de vade-mecum et de foires aux questions, dont les réponses deviennent autant de directives dictées depuis la rue de Grenelle. Vous n'avez pas su, vous n'avez pas pu, desserrer l'étau qui étouffe le dernier système éducatif centralisé et bureaucratisé d'Europe. On est bien loin d'un ministère qui se recentrerait sur l'essentiel, d'un ministre qui n'écrirait aux professeurs que lorsque c'est indispensable, laissant la main aux recteurs chaque fois qu'il n'est pas impératif que les décisions soient prises à Paris. En conclusion, il est indéniable que les réformes engagées partaient pour la plupart d'intentions louables. Mais, finalement, le bilan, en demi-teinte, apparaît bien insuffisant au regard de l'ampleur de la crise de l'école et de toute une série de modes de fonctionnement anciens, qui s'essoufflaient, et s'essoufflent encore, inlassablement. Je veux bien concéder que la crise sanitaire a largement perturbé votre action. Mais il est bien difficile de dire qu'aujourd'hui l'école se porte mieux qu'il y a cinq ans. L'engagement des professeurs n'est pas en cause. C'est un problème d'organisation comme d'autres avant vous, au nom de l'égalitarisme, confondu avec la recherche de l'équité, vous avez privilégié le saupoudrage et bridé les initiatives. Comme celles d'autres avant vous, vos réformes se sont enlisées. Contre cet enlisement, il n'y a qu'un antidote : plus de liberté pour les écoles et les établissements, et une nouvelle conception du métier de professeur et de sa place dans la société.

Celui qui s'ouvre ce soir sera, j'en suis certain, l'occasion de dresser un tableau des faiblesses et des lacunes de notre système éducatif, mais aussi de ses atouts et des raisons d'espérer, pour répondre enfin aux enjeux de l'école de demain. La parole est à M. le ministre.

tous ceux qui y parvenaient étaient dans la concession vis-à-vis des organisations syndicales ou de tous les groupes de pression. Vous considérez apparemment, monsieur le sénateur, que je n'ai pas suffisamment été soumis à cette pression ... L'important, aujourd'hui, aujourd'hui, est de voir que des sillons ont été creusés. Vous le savez parfaitement, monsieur le sénateur : en matière éducative, il faut savoir semer des graines. Je ne prétends pas que nous sommes à l'heure des moissons ; je prétends que nous sommes au moins à l'heure des bourgeons. Et ces bourgeons sont là, devant nous : ils sont réels.

le dernier classement international date de 2018. Il émane du PISA et concerne des élèves de quinze ans. Oui, quand je suis arrivé, la situation n'était pas bonne ; oui, le lycée était à bout de souffle. cela faisait 20 ans qu'on parlait de la réforme nécessaire du baccalauréat. Oui, quand je suis arrivé, le niveau de mathématiques était très faible, et il n'y avait qu'une faible proportion d'élèves issus de la filière S dans les filières scientifiques,

Quand je suis arrivé, la rémunération des enseignants n'était pas à la hauteur. Certes, il reste encore beaucoup à faire, j'y reviendrai, mais nous avons procédé à des augmentations. Il ne s'agit Il ne s'agit pas de dire que rien n'avait été fait avant nous, bien entendu. Je pense notamment à la politique d'éducation prioritaire, qui a franchi des étapes importantes depuis les années 1980, ou à la politique de l'école inclusive, qui a commencé avec Jacques Chirac, et à laquelle nous avons fait faire un nouveau pas très important. Je ne ferai pas, pour ma part, une sorte de procès manichéen à tous ceux qui m'ont précédé. Mais il est certain certain que la situation était difficile et que les changements à faire étaient nombreux. Les priorités ont été indiquées d'emblée : la réforme de l'école primaire, d'abord, puis l'évolution de l'enseignement professionnel, enfin, la réforme du lycée général et technologique. Autant de totems auxquels personne ne s'était attaqué comme cette majorité l'a fait. Les objectifs étaient clairs, aussi : l'élévation du niveau général et la lutte contre les inégalités. Non, monsieur le sénateur Brisson,

L'enseignement public est, bien évidemment, délivré en français. Cependant, de très nombreux élèves accueillis dans les classes ne parlent que le créole haïtien ou l'espagnol. Ainsi l'enseignement scolaire à Saint-Martin est-il très compliqué, car le multilinguisme y est particulièrement prononcé. En conséquence, les enseignants sont confrontés à des classes très hétérogènes, tant du point de vue linguistique que par les différences de milieux socioculturels. Le rectorat de la Guadeloupe, tout comme les services de l'éducation nationale de Saint-Martin, a pleinement conscience de ces enjeux, puisqu'un enseignement bilingue y est dispensé à quelques élèves. C'est ainsi qu'à la rentrée 2021, on comptait dans le premier degré, de la moyenne section au CM1, 30 classes

Ces initiatives portent leurs fruits. Elles doivent donc être confortées et renforcées, afin de lutter notamment contre le très fort taux d'échec scolaire que nous connaissons malheureusement.

un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter l'apprentissage de la langue française. Les élus du conseil territorial ont déjà délibéré en ce sens à l'unanimité. Pouvons-nous compter sur un accompagnement de l'État, qui pourrait permettre la généralisation de l'enseignement bilingue sur l'ensemble du territoire de Saint-Martin ? La parole

Medef s'inquiète en effet de voir s'évaporer un vivier d'ingénieurs et, j'ajouterai, de femmes ingénieures. La réforme du lycée que vous avez conduite, avec la suppression des mathématiques du tronc commun de première et terminale générale, a eu de fâcheuses conséquences : les mathématiques ne sont plus une matière obligatoire, mais une spécialité de six heures par semaine en terminale pour celles et ceux qui la choisissent, soit 37 % seulement des élèves.

Nous courons donc un risque de pénurie d'ingénieurs, notamment d'ingénieurs informatiques. Si cette discipline attire moins les élèves, c'est aussi par manque d'information sur les attentes de l'enseignement supérieur et par peur de se voir sanctionné par le système Parcoursup. Autre alerte : après des décennies d'efforts pour arriver à un quasi-équilibre entre garçons et filles dans les filières scientifiques, le ratio s'est écroulé en seulement deux années. Cette spécialité est devenue excluante. Nous assistons à un retour des stéréotypes de genre, qui aura pour conséquence l'accentuation des inégalités femmes-hommes, pourtant supposée être- rappelons-le -la grande cause du quinquennat. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'il faudrait renforcer le rôle et le nombre- qui est insuffisant -des conseillers d'orientation psychologues en collège et en lycée, qui sont actuellement en moyenne d'un pour 1 500 élèves ? Enfin, et surtout, comment comptez-vous réorienter votre réforme, conspuée de toutes parts, pour répondre à cette baisse de niveau en mathématiques, qui creuse des inégalités sociales et de genre ? Très bien

des mesures en faveur d'une école de proximité, qui tourne le dos à une gestion « comptable ». Allez-vous entendre les protestations contre les fermetures de classe en éducation prioritaire,

Comptez-vous ouvrir plus de postes pour la prochaine session des concours ? Les heures supplémentaires ne remplacent pas les postes, tous les chiffres en attestent. Quant aux accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), nous en manquons encore terriblement et leur statut reste excessivement précaire. vient par ailleurs de les transférer subrepticement aux collectivités, notamment sur les temps de restauration. Comptez-vous assumer la rémunération complète des AESH ? Très bien

Aucun autre mandat n'a donné lieu à une telle augmentation ! À l'école primaire, où nous avons concentré les augmentations de moyens- et j'en suis fier -, plus de 11 000 postes ont

sur sa politique menée depuis cinq ans. C'est la réalité des chiffres ! Je remarque qu'il y a une dizaine de jours- un mois tout au plus -toute la communauté éducative était réunie dans la rue dans une mobilisation absolument inédite. Vos chiffres disent certainement des choses, monsieur le ministre,

du niveau des lycéens en la matière, ainsi qu'un faible taux de féminisation dans les filières scientifiques et techniques. La réforme du lycée de 2019 a entraîné une chute historique du nombre d'élèves suivant des cours de mathématiques en première et en terminale. Une donnée illustre à elle seule les écueils de cette réforme : de 2018 à 2020, le nombre d'heures de cours dispensées en mathématiques a diminué de 18 %. Pour corriger sa copie, le Gouvernement a lancé, la semaine dernière, une consultation sur le sort des mathématiques au lycée. En cette période électorale, je m'interroge avec bienveillance, monsieur le ministre, sur le tempo de cette annonce pour le moins tardive. Nous attendrons, malgré tout, des garanties concrètes sur ce qui pourrait en résulter. Enfin, permettez-moi d'aborder un second point, qui conditionne en bonne partie l'avenir de nos futurs étudiants. En février 2020, la Cour des comptes soulignait que 65 % des proviseurs et 85 % des professeurs principaux n'avaient reçu aucune formation spécifique pour exercer leur mission d'orientation. Monsieur le ministre, mes questions sont simples : quelles garanties comptez-vous donner aux enseignants, aux parents d'élèves et aux lycéens quant à l'avenir des mathématiques dans le tronc commun ? Que comptez-vous faire pour renforcer le temps de formation des professeurs principaux afin d'améliorer l'orientation de nos jeunes générations ? La parole est à M. le ministre. Il est

part de PIB supérieure à nombre de nos voisins- Allemagne en tête -et, cependant, un montant consacré par élève inférieur ; plus d'heures consacrées aux fondamentaux et pourtant inégalité sociale aggravée

Mais l'éducation nationale, comme nous avons la prétention de l'appeler, ne se résume pas à l'instruction et à la transmission des savoirs. Trois mondes cohabitent trop hermétiquement : l'école, la famille et la rue, où hélas ! certains enfants passent trop de temps. Un comportement inadapté en milieu scolaire trouve parfois son inspiration dans la rue, où il doit être encadré. Les difficultés d'acquisition nécessitent un soutien familial qu'il faut accompagner. De façon plus évidente encore, la

Il n'y a pas de pathologies spécifiques à l'école. Le dépistage du handicap, qu'il soit auditif, visuel ou d'attention, est nécessaire à l'école comme en famille ou dans la vie en général. Quel sens donner au travail des assistantes sociales si celles-ci ne peuvent pas coordonner leurs interventions dans les familles et à l'école ? Il en est de même pour les surveillants scolaires, les intervenants périscolaires et les éducateurs de rue.

Ce choix est motivé avant tout par des considérations de vie sociale et familiale et il a été arrêté en fonction des contraintes et des préférences des adultes, mais il reste en totale inadéquation avec les besoins des enfants. Pourtant, de nombreuses études de chronobiologistes montrent que ce type de fonctionnement s'accompagne d'une baisse du niveau de performance, en particulier chez les enfants des milieux défavorisés, qui ne bénéficient pas de structures périscolaires et extrascolaires, de sorte qu'ils se retrouvent malheureusement trop souvent livrés à eux-mêmes. Il est désormais avéré que les apprentissages se font mieux pendant les matinées. Le fait d'en supprimer une par semaine, soit trente-six par an, est évidemment dommageable pour la réussite de nombreux enfants de nos écoles.

de jours d'école pour un nombre total d'heures plus élevé en moyenne. Il y a là une contradiction. Le précédent gouvernement en avait tiré des enseignements en proposant d'abandonner la semaine de quatre jours, telle qu'elle avait été imposée par le Gouvernement en 2008, d'introduire une neuvième demi-journée plus favorable au travail scolaire et à l'épanouissement des enfants. Toutefois, l'expérience n'aura pas assez duré pour qu'on en mesure les bienfaits et les nombreux égoïsmes autour de l'école et dans l'école auront bientôt raison de cet allongement bénéfique de la semaine avec cinq matinées favorables aux apprentissages. Ajoutons à cela la disparition quasi générale des activités culturelles et sportives, faute de temps, dans une semaine désormais concentrée sur les disciplines de base. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire de rouvrir le dossier des rythmes scolaires dans nos écoles ?

l'ouverture de 1 500 places en internat d'excellence. Cet objectif sera-t-il atteint ? Pouvez-vous nous dire où en est l'installation de ces internats dans les territoires ? La parole

toute une série de références que nous avons créées. Oui, les savoirs fondamentaux se sont consolidés pendant ce mandat, tout particulièrement dans les réseaux d'éducation prioritaire ; c'est aussi dans l'ensemble du système éducatif français que l'on observe ces améliorations.

Il met en exergue un déclin général du niveau des études. En effet, nous sommes classés au 23 rang pour la lecture et la compréhension de texte. Ne parlons pas de l'effondrement du niveau en français, en orthographe, en histoire-géographie ou en langues vivantes la France se situe en dessous de la moyenne de l'Union européenne et des pays de l'OCDE, notamment en mathématiques. Les réformes se sont succédé à un rythme soutenu depuis plusieurs décennies, mais leur avons-nous laissé le temps de déployer tous leurs effets avant de réformer de nouveau ? Il faut parfois des années pour pouvoir dresser un bilan. Cette frénésie législative complique le quotidien des enseignants. Force est de constater que leur métier est de moins en moins attractif. Le mauvais rendement des concours, dû au manque de candidats dans les disciplines majeures, et les vagues de démissions de ces dernières années sont révélateurs.

Le système éducatif des pays nordiques repose en grande partie sur l'autonomie des professeurs, notamment pour organiser leur travail. Les classes sont moins nombreuses, ce qui facilite une meilleure adaptation des méthodes. Ce système semble faire ses preuves puisque les pays nordiques sont en tête des classements PISA. Monsieur le ministre, l'inquiétude est à la mesure de l'enjeu. Quelles sont nos marges de manoeuvre sur le sujet ? Pourquoi ne pas nous inspirer davantage du système nordique qui fonctionne mieux ?

En français et en mathématiques, il y a un plan qui s'accompagne de références pédagogiques élaborées par un conseil scientifique de l'éducation nationale. Il y a aussi le dédoublement des classes, qui est une mesure phare, les évaluations de début d'année, qui nous permettent d'être le seul pays au monde à avoir une

Ces chiffres révèlent une tendance de fond : l'éducation nationale aura de plus en plus de mal à susciter des vocations. Comment en sommes-nous arrivés là ? Il est évident que la question des salaires est importante. Après un début de carrière à 1 600 euros net, un enseignant qui a atteint dix ans d'ancienneté perçoit un traitement inférieur de 15 % à la moyenne de l'OCDE. Monsieur le ministre, qu'en est-il de la hausse des salaires promise ? Un autre facteur d'explication se trouve dans l'obligation de posséder un bac+5 pour passer le concours d'enseignant alors qu'une licence suffisait auparavant. Enfin, les conditions de travail, monsieur le ministre, ne sont guère de nature à motiver les futurs enseignants. Il est de notoriété publique que nombre d'entre eux ne se sentent plus soutenus par leur hiérarchie en cas de difficultés avec leurs élèves.

Le métier ne suscite plus vraiment l'enthousiasme des diplômés. Monsieur le ministre, le Gouvernement a-t-il conscience de ce phénomène ? Comptez-vous agir pour l'enrayer avant qu'il ne prenne trop d'ampleur ?

hausse inédite du budget de l'éducation nationale, soit 13 % au cours de ce quinquennat, ainsi qu'une augmentation inédite du salaire des jeunes professeurs. Vous avez évoqué le chiffre de 1 600 euros, très obsolète

J'ai tenu des propos très clairs, dès ma prise de fonction, sur la défense des professeurs et je n'ai pas changé d'un iota sur cette question. Vous avez raison de faire un entre

par exemple, des parents d'élèves qui ont été violents verbalement ou physiquement avec des professeurs. J'ai été d'une rigueur d'airain sur ce sujet. Tout fait signalé fait l'objet de poursuites. J'en constate tous les jours. Je regrette comme vous le phénomène de société qui accroît l'agressivité.

de La Provôté. Monsieur le ministre, ma question porte sur l'éducation prioritaire, l'expérimentation en cours des contrats locaux d'accompagnement et les territoires éducatifs ruraux. expérimentation a deux objectifs : améliorer les dispositifs existants, qui ont beaucoup apporté à l'édifice, mais qui n'ont pas obtenu des résultats performants, et davantage prendre en compte les inégalités territoriales. Ainsi, depuis la rentrée 2021, 172 écoles, collèges et lycées des académies de Nantes, Lille et Marseille sont concernés et un contrat a introduit la progressivité dans l'allocation des moyens, et ce pour une durée de trois ans. Ces objectifs avaient été mis en avant dans le rapport sénatorial rendu en octobre 2019 par nos collègues Laurent Lafon et Jean-Yves Roux au nom de la mission d'information sur les nouveaux territoires de l'éducation une meilleure équité territoriale est nécessaire. L'éducation prioritaire ne s'éteint pas à la couronne périurbaine de chaque ville et les territoires ruraux ont aussi des besoins en la matière. Or, depuis sa création, il y a quarante ans, l'éducation prioritaire fondée sur les inégalités sociales s'est concentrée sur les grands quartiers urbains. Quel que soit le territoire, l'objectif est bien finalement identique : c'est la réussite des élèves par des moyens différenciés et adaptés. Monsieur le ministre, cela fait six mois que dure l'expérimentation. Il était prévu de l'élargir à d'autres académies en cas de bons résultats ou si le dispositif démontrait son efficacité.

de contractualisation pour faire ce que nous avons appelé des « alliances éducatives ». Ce dispositif répond à plusieurs questions qui ont été posées jusqu'à présent. Un peu comme dans l'esprit des cités éducatives, l'objectif est d'avoir un impact sur les facteurs extrascolaires, par exemple les activités sportives et culturelles des élèves en milieu rural, en plus de leur activité scolaire. Il existe donc désormais un cadre qui va de pair avec la revitalisation des internats d'excellence et la politique en faveur des écoles rurales. Il doit permettre de développer une véritable politique d'appui à ces territoires éducatifs ruraux. Il s'inscrit également dans le même objectif que l'extension cordées de la réussite aux collèges ruraux depuis la rentrée 2020 : quelque 20 000 collégiens sont accompagnés dans ce cadre en territoire rural.

En d'autres termes, au lycée, l'apprentissage des mathématiques est devenu à double vitesse, accentuant les inégalités sociales et de genre. Pour preuve, en 2019, les filles représentaient 47,7 % des effectifs en en 2021, elles ne sont plus que 39,8 % à avoir choisi la spécialité « maths », soit au-dessous du niveau de 1994. Ce décrochage soudain et massif est une régression. D'ailleurs, les instituts de recherche, les associations et aussi les collectifs de professeurs de mathématiques ne s'y trompent pas : ils vous ont alerté dans une missive et ils pointent même le caractère édifiant de ce décrochage. Cette rupture a des incidences préjudiciables en matière de débouchés. Mécaniquement, se pose le problème de l'accès aux filières scientifiques, économiques et numériques, lesquelles constituent la priorité du plan France 2030 et concentrent la majorité des investissements. Autrement dit, la place de la discipline mathématique conditionne le succès de la France dans ces filières, érigées comme prioritaires. Rappelons qu'il manque 5 000 ingénieurs par an. Aujourd'hui, cette inadéquation est une question éminemment politique. Le recrutement et la formation des enseignants, l'attractivité des carrières, la pédagogie à l'oeuvre en classe et le travail sur les représentations constituent autant de sujets à traiter.

pour sécuriser leur saut dans le nouvel univers de Parcoursup, les élèves doivent dorénavant s'appuyer sur les conseils de leurs professeurs principaux. La réforme du lycée a ainsi érigé l'accompagnement à l'orientation en impératif,

notamment dans les universités. Force est de constater que les actions mises en place sont très hétérogènes- elles dépendent des établissements et des équipes -et manquent clairement de lisibilité et de cohérence.

la crise sanitaire a changé la donne : les salons de l'orientation se sont transformés en visites et conférences virtuelles, parfois déroutantes pour les lycéens. Monsieur le ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour que les lycéens, déjà malmenés par la crise sanitaire, ne manquent pas d'ambition, simplement à cause d'une méconnaissance des formations existantes ?

Certes, plusieurs mesures issues du Grenelle de l'éducation constituent des avancées appréciables pour diverses catégories de personnel, mais elles ne sauraient masquer le refus du Gouvernement d'ouvrir la question centrale de la revalorisation du point d'indice, alors qu'un contexte inflationniste s'installe durablement.

le même temps, il convient d'évoquer la situation des AESH et des APSH, qui accomplissent des missions essentielles au sein de l'école, dont le rôle inclusif

ou une France ayant préservé un cadre de vie diversifié et respectant ses traditions et les attentes des Français, en leur laissant le choix de leur lieu de vie

La prise en charge de la difficulté scolaire tout au long du parcours des élèves est bien installée dans l'établissement. [ ...] Une amélioration des résultats au diplôme national du brevet est perceptible depuis trois ans. [ ...] Les élèves semblent mieux comprendre et vivre les transitions inhérentes au parcours scolaire. » Forte de ce diagnostic optimiste et encourageant, l'expérimentation menée sur le territoire de Jussey s'est poursuivie et entre désormais dans sa quatrième année. Si la crise sanitaire a retardé l'objectivation des résultats, il n'en demeure pas moins que l'école du socle, de l'avis de la communauté éducative, produit des résultats toujours aussi prometteurs. Les élèves en milieu rural sont moins préoccupés par le changement de degré scolaire. Leurs chances de réussite sont donc optimisées. Nous constatons également que l'école du socle a ouvert les portes d'une acculturation entre les enseignants, de la petite section de maternelle à la classe de

quand et comment prévoyez-vous de consacrer les écoles du socle ? La

le bilan de la politique éducative française est sévère. Pourtant, je me refuse à la perspective de voir notre pays condamné au déclin de son école. Il apparaît ainsi clairement que la faiblesse de notre système éducatif tient au manque d'une stratégie globale et de long terme. L'école est une institution centrale au coeur de la promesse républicaine d'égalité des chances. Or celle-ci reste aujourd'hui lettre morte. Pis encore, les travaux du centre de recherches politiques de Sciences Po montrent que l'effondrement de la confiance des Français dans la démocratie s'explique largement par cette crise de la méritocratie républicaine.

Que dire de cette étude montrant que la moitié des différences de croissance entre les pays s'explique par le différentiel de niveau en mathématiques et en sciences ? Les performances de la France en la matière sont très décevantes.

outil de consolidation de notre société, de partage de valeurs et de construction de l'avenir. Je voudrais remercier le groupe Les Républicains d'avoir accepté la demande de Max Brisson d'ouvrir ce débat.

des candidats à cet enseignement est trop faible, et les concours en subissent évidemment les conséquences. Par ailleurs, nos professeurs des écoles sont essentiellement des littéraires,

nos instituts de recherche et nos entreprises, nos capacités d'innovation en santé souffrent à présent d'un certain retard par rapport à celles de nos voisins. La France a largement sous-estimé certaines tendances lourdes, dont l'effacement des frontières entre recherche fondamentale et recherche clinique et appliquée, le besoin d'investissements massifs pour prendre le virage des biotechnologies, ou encore la délocalisation des capacités de production en principes actifs. L'indépendance sanitaire française en a été sérieusement entamée. Les difficultés que notre pays a éprouvées dans la production d'un vaccin contre la covid-19, en comparaison avec les États-Unis, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, sont symptomatiques de cette nouvelle donne paradoxale, faite d'excellence de la recherche « à la française » et de corsetage manifeste de ses potentialités. Résoudre cette tension est un impératif : il y va de l'accès des patients aux thérapies les plus susceptibles de les soigner. c'est ce à quoi s'emploie la proposition de loi que je vous présente ce soir. Elle découle de la fusion de deux précédentes propositions qu'Annie Delmont-Koropoulis et moi-même avions rédigées séparément, en 2019 et 2020. Elle est quelque peu technique, j'en conviens, mais peut constituer une réelle avancée pour les acteurs de la recherche et pour les patients, ce qui est le plus important. texte articule la défense de grands objectifs, comme la souveraineté sanitaire et le développement de la médecine personnalisée, avec la mise en oeuvre de solutions concrètes pour fluidifier les procédures d'évaluation des recherches et permettre aux acteurs de l'écosystème de l'innovation en santé de produire, sans obstacle superflu, les traitements innovants les plus adéquats pour les patients. Les dysfonctionnements sont, pour certains, identifiés depuis assez longtemps. La question de l'accès précoce est une préoccupation ancienne et constante de notre commission. Dans un rapport que j'avais cosigné avec Yves Daudigny et Véronique Guillotin en juin 2018, en préparation du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS), la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) avait évalué le modèle français de l'accès précoce en cherchant à objectiver les conditions et les délais de mise à disposition des thérapies innovantes à chacune des étapes, des essais cliniques à la commercialisation des médicaments après leur autorisation de mise sur le marché (AMM), en passant par le système spécifique des autorisations temporaires d'utilisation (ATU). éléments ont été précisés dans le rapport coécrit par Annie Delmont-Koropoulis, rapporteure de cette proposition de loi, et Véronique Guillotin dans le cadre du CSIS de 2021, qui a fourni en juin dernier un état des lieux actualisé de la situation, assorti de recommandations opérationnelles nouvelles. Certaines avancées proposées par ces rapports ont été réalisées, comme les extensions d'indications. D'autres devraient être mises en oeuvre prochainement par le Gouvernement, comme la création d'une agence de l'innovation en santé. Peut-être le secrétaire d'État nous en dira-t-il davantage sur le calendrier de sa création, annoncée en décembre dernier par le Premier ministre. D'autres dysfonctionnements font précisément l'objet du présent texte. Nos deux collègues rapporteures proposaient ainsi de moderniser le fonctionnement des comités de protection des personnes, les CPP. Ces comités, chargés d'émettre un avis préalable sur les conditions de validité de toute recherche impliquant la personne humaine, sont aujourd'hui surchargés. Cet engorgement retarde les essais cliniques indispensables à l'élaboration de nouveaux traitements. L'article 6 s'attaque tout particulièrement à ce sujet et propose une solution originale pour externaliser les dossiers de recherches non interventionnelles, qui sont les dossiers en plus forte croissance, vers d'autres acteurs. Il est en cela conforté par les articles 4, 5, 8 et 9, qui visent à améliorer le fonctionnement et à renforcer l'attractivité de ces comités de protection des personnes, à organiser leur évaluation et à favoriser les bonnes pratiques, ainsi qu'à renforcer la prévention des conflits d'intérêts par la création d'un déontologue au sein de la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine. Il s'agit aussi de donner corps à la notion de souveraineté et de sécurité sanitaire, que la proposition de loi range parmi les objectifs des stratégies nationales de recherche et de santé, avec l'amélioration de la qualité de vie. L'autre grand enjeu de cette proposition de loi est l'accès des patients aux innovations. Le forfait diagnostic cancer prévu par l'article 14 et la détermination, par l'article 16, d'un critère nouveau de « valeur thérapeutique relative » sont autant de dispositions qui entendent favoriser l'accès des patients aux fruits de l'innovation médicale. La facilitation des essais cliniques en ambulatoire, l'organisation du transport sanitaire des enfants atteints de pathologies rares vers les centres spécialisés y contribuent de façon plus indirecte, mais tout aussi importante. le texte introduit dans la loi la définition de la médecine personnalisée. Certains la connaissent sous le terme de « médecine de précision », « médecine 4P » ou Son développement s'appuierait sur la recherche appliquée en santé, également définie par l'article 12, ainsi que sur des volets spécifiques au sein de la stratégie nationale de santé et de la stratégie nationale de recherche, comme le prévoit l'article 13. À la fluidification de l'évaluation des recherches, à la facilitation de l'accès des patients à l'innovation, à la consécration des objectifs de souveraineté sanitaire et de développement de la médecine personnalisée, s'ajoutent enfin quelques dispositions sur la problématique des données personnelles de santé. L'accès à ces données d'une incroyable richesse doit être facilité pour mieux comprendre les effets d'un traitement. C'est tout l'enjeu, notamment, de l'exploitation des données en vie réelle, sur lesquelles la Haute Autorité de santé doit s'appuyer plus systématiquement. L'accès aux données de santé doit toutefois faire l'objet d'un encadrement équilibré : la confiance de nos concitoyens dans le système national des données de santé (SNDS) est effectivement indispensable pour permettre à ce dernier de déployer son plein potentiel au bénéfice des patients. La sécurisation du stockage des données personnelles de santé au niveau européen, visée par l'article 22, est un moyen déterminant du renforcement de cette confiance. Anticipant quelque peu sur la mission d'information relative aux données de santé que la commission des affaires sociales lancera très prochainement, je saisis d'ailleurs l'occasion fournie par l'examen de cette proposition de loi pour vous demander, monsieur le secrétaire d'État, davantage d'explications sur les conditions dans lesquelles le contrat de prestation liant liant Microsoft et la plateforme des données de santé a été conclu en avril 2020. Où en sont, par ailleurs, la recherche et le développement des solutions techniques de substitution de niveau européen pour héberger et gérer les données personnelles de santé Il ne paraît pas possible de se satisfaire de la situation actuelle, qui est, il faut bien le dire, assez bancale. Cette proposition de loi me semble offrir un arsenal de mesures cohérent et assez large pour développer l'innovation en santé sur notre territoire. Je voudrais enfin remercier la rapporteure, Annie Delmont-Koropoulis, qui a conduit un travail de consultation de grande ampleur sur ce texte et l'a profondément amélioré, conformément aux intentions de son auteure, un souci permanent de prise en compte des réalités de terrain. Elle est allée jusqu'à proposer des solutions assez audacieuses pour faire sauter les derniers verrous- je songe au désengorgement des comités de protection des personnes ou à la création de CPP spécialisés.

en 2019 et en 2020, ainsi que celles qui sont issues des derniers travaux de la commission, notamment le rapport que j'ai coécrit avec Véronique Guillotin dans le cadre du CSIS de 2021. J'ai en outre auditionné, pour l'occasion, près d'une soixantaine de personnes, reflétant toute la richesse de l'écosystème de la recherche en santé : acteurs de la recherche académique, industriels du médicament, spécialistes des traitements innovants en oncologie ou en pédiatrie, autorités de régulation, entrepreneurs des biotechs, acteurs de l'évaluation éthique de la recherche. Il s'agissait pour moi de solliciter les vues les plus larges sur ce sujet d'importance majeure, pour les patients d'abord, pour le rang de la France dans la compétition scientifique et industrielle ensuite. Le premier volet de ce texte vise à améliorer le système d'évaluation éthique des recherches conduites dans le domaine de la santé. En effet, toute recherche impliquant la personne humaine doit faire l'objet d'un avis favorable d'un comité de protection des personnes. Or ces instances sont mal équipées pour absorber la charge de travail qui leur revient. D'où les solutions proposées par le texte : mieux les équiper et alléger cette charge de travail. L'article 3 visait ainsi, afin de garantir aux comités les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leurs missions, à les rattacher systématiquement à un La commission a proposé d'élargir cette possibilité aux centres hospitaliers et aux établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif- qui peuvent être, par exemple, des centres de lutte contre le cancer. Elle a également proposé que certains CPP soient spécialisés en pédiatrie et en maladies rares, car ce sont des compétences spécifiques, dont la bonne identification contribuera à soutenir le développement des recherches. L'article 8 prévoit la valorisation de la participation aux travaux des CPP dans la carrière des universitaires et praticiens hospitaliers, afin de remédier au déficit d'attractivité de ces activités, aujourd'hui faiblement indemnisées et exercées pour l'essentiel par des passionnés. L'allégement de la charge de travail des CPP fait l'objet de l'article 6. Plus d'un tiers des demandes de recherche soumis aux CPP pour évaluation sont des recherches non interventionnelles. Il s'agit de la

le nombre de RIPH 3 a vocation à croître encore. Dans notre rapport, Véronique Guillotin et moi-même proposions de transférer ces dossiers à un comité d'éthique spécialisé. L'Inspection générale Les auditions m'ont toutefois conduite à reconsidérer le problème. Peu d'interlocuteurs semblent croire à la solution du comité unique spécialisé, pour des raisons tenant à son volume d'activité attendu et au risque de concentration des conflits d'intérêts.

La commission a finalement accepté de suivre ma proposition consistant à décharger les CPP des RIPH 3 en faisant appel aux comités d'éthique de la recherche (CER) qui existent déjà. Ces comités, aujourd'hui consultatifs et logés dans les universités, examinent les recherches n'impliquant pas la personne humaine au sens de la loi Jardé, qui peuvent concerner la santé, mais aussi les sciences de l'homme. S'il arrive que des membres de CER soient aussi membres de CPP, on peut dire, je crois, que les deux mondes s'ignorent largement. Qu'est-ce qui empêche pourtant d'imaginer leur convergence, jusqu'au partage, dans des conditions ne privant pas les CPP de leur compétence, d'une matière commune, laquelle a pour principal critère de définition d'être sans risque pour les personnes se prêtant à la recherche Cela exigera, certes, de porter les CER au niveau de compétences qui est exigé pour ce type de recherches. Or il se trouve que conférer une base légale et mieux encadrer la création, le fonctionnement et l'évaluation des CER, c'est précisément l'objet de l'article 9.

constituer un référentiel commun, établir un annuaire des experts mobilisables, proposer des formations et abriter un déontologue chargé de prévenir les conflits d'intérêts. Toujours afin de faciliter et mieux encadrer la recherche, l'article 1 précise les dispositions relatives aux essais cliniques en ambulatoire, rend possible le recours à la télémédecine lorsque les patients sont suivis à domicile et tâche de remédier au problème du transport des enfants atteints de pathologies rares vers les centres spécialisés, qui sont donc peu nombreux et mal répartis, où les essais cliniques peuvent être conduits. Le deuxième volet de ce texte vise à soutenir la recherche dans le domaine de la médecine personnalisée. Les articles 11 à 13 à faire du développement de la médecine personnalisée un objectif commun aux politiques de recherche et de santé publique. L'article 11 prévoit que la politique nationale de recherche et la recherche publique contribuent au renforcement de la souveraineté et de la sécurité sanitaire, ainsi que de l'amélioration de la qualité de vie. Pour améliorer la qualité de prise en charge, rangée par l'article 12 parmi les objectifs de la politique de santé, la médecine personnalisée, désormais définie comme l'adaptation des actions de prévention et des stratégies diagnostiques et thérapeutiques aux spécificités du patient et de l'affection, serait selon moi un puissant adjuvant. consiste à favoriser l'accès des patients à l'innovation. L'article 14 introduit un mécanisme original visant à mieux prendre en charge le diagnostic d'un cancer. De tels actes sont aujourd'hui financés

avec Dominique Stoppa-Lyonnet, professeure de génétique et ancienne membre du Comité consultatif national d'éthique, cet article consiste à prendre en charge forfaitairement la recherche de biomarqueurs diagnostiques, pronostiques ou théranostiques pour tout nouveau cancer diagnostiqué chez un patient. L'article 15 confie à la Haute Autorité de santé une mission de veille et de prospective, que la future Agence de l'innovation en santé exercera peut-être, mais qu'il n'est pas inutile, en attendant, d'inscrire dans la loi. En outre, il assouplit légèrement l'organisation de la Haute Autorité. Les articles 16 et 18 visent à favoriser l'accès des patients aux médicaments innovants. Le premier prévoit, à titre expérimental, que le Comité économique des produits de santé (CEPS) pourra fonder le prix d'un médicament innovant, dont l'amélioration du service médical rendu est par hypothèse difficile à mesurer par comparaison avec un autre, sur un critère nouveau, celui de sa « valeur thérapeutique relative », qui serait soumis à des réévaluations périodiques en fonction des données de vie réelle collectées. La dernière partie du texte est relative aux données de santé. Les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou les exploitants d'un traitement peuvent avoir besoin, pour évaluer son efficacité en vie réelle, d'accéder aux données de santé du SNDS. L'article 20 vise à mieux encadrer cet accès et à le conditionner à la remise annuelle d'une étude évaluant les effets de la prescription des produits, ainsi qu'à la validation d'un protocole de recherche par le comité compétent. Les articles 21 et 22, enfin, visent à renforcer les garanties des citoyens patients quant à l'usage de leurs données personnelles de santé. L'article 21 interdit l'usage de ces données par les organismes complémentaires à des fins de sélection des risques. L'article 22 tend à sécuriser le stockage des données en santé en réservant leur hébergement et leur gestion à des opérateurs relevant exclusivement de la juridiction de l'Union européenne. Certes, il n'existe pas encore de solution technique souveraine à même de remplacer Microsoft Azure, l'outil auquel la plateforme des données de santé a recouru pour héberger et gérer et gérer les données de santé du SNDS. Toutefois, les risques sont réels et ils peuvent saper la confiance de nos concitoyens dans le SNDS, entravant ainsi le plein déploiement de ses capacités, en particulier au bénéfice de l'innovation en santé. Je salue à ce propos l'ouverture de l'espace numérique de santé, indispensable pour améliorer le suivi des patients, ainsi que la coordination entre les médecins traitants et les spécialistes. Vous le voyez, mes chers collègues, ce texte s'efforce, dans un format réduit, de lever un certain nombre de freins à l'innovation en santé, dans le souci de soutenir l'ensemble de l'écosystème. Puisse-t-il bénéficier de la navette pour être amélioré et profiter à la recherche et à notre pays dans son ensemble !

Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales, chère Catherine Deroche, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi que vous vous apprêtez à examiner a pour objet de renforcer l'évaluation éthique de la recherche en santé et d'améliorer les conditions d'accès aux thérapies innovantes- autant d'objectifs que nous partageons pleinement. Je tiens à saluer l'investissement de la commission

Concernant tout d'abord les recherches impliquant la personne humaine, permettez-moi de rappeler que l'une des priorités du Gouvernement dans le cadre du plan Innovation Santé 2030 est précisément de renforcer l'attractivité de la France en matière de recherche. Notre objectif est d'augmenter le nombre d'essais cliniques et le nombre de patients inclus, notamment par une réduction significative des délais d'autorisation, tout en conservant évidemment un haut niveau de qualité méthodologique et éthique. Pour y parvenir, le Gouvernement a engagé de nombreuses actions en vue de réduire drastiquement les délais d'évaluation des projets de recherche et de préparer l'entrée en vigueur de règlements européens. Les moyens des comités de protection des personnes (CPP) ont ainsi été renforcés, grâce notamment à une hausse de 5 millions d'euros des budgets consacrés à l'évaluation éthique des produits de santé, au recrutement de renforts administratifs, à la revalorisation des indemnités des membres ou encore à la mise en place de nouveaux cycles de formation. Le ministère a par ailleurs mis en place une plateforme de support et d'animation du réseau des comités pour harmoniser leurs pratiques. Un pôle a aussi été créé à la fin du mois de janvier dernier pour renforcer leur coordination. Toutes ces réformes sont nécessaires au regard des évolutions réglementaires européennes, qui prévoient des délais d'évaluation plus courts, et du fait que le silence des comités vaut avis favorable, ce qui rend indispensable le respect des délais impartis.

Le renforcement des moyens des CPP ne leur permettra toutefois pas d'évaluer dans les délais réglementaires l'ensemble des projets de recherche impliquant la personne humaine soumis chaque année. Il y a trop de recherches déposées pour les 39 comités. Il faut donc créer d'autres structures et élargir le vivier de recrutement des personnes volontaires.

proposition de loi prévoit de confier à d'autres structures la mission d'évaluation des recherches non interventionnelles. Une telle évolution semble à terme indispensable

l'objet d'une concertation avec les acteurs du secteur, nous semblent constituer le bon équilibre. Elles visent à confier l'évaluation des recherches non interventionnelles à des comités d'éthiques locaux de la recherche, créés par des établissements de santé et coordonnés par une commission nationale. Plusieurs autres dispositions figurant dans cette proposition de loi nous semblent intéressantes, notamment celles qui portent sur la recherche en ambulatoire, la pérennisation d'une procédure d'évaluation accélérée des recherches en cas d'urgence sanitaire ou la valorisation de l'activité de rapporteur de projets de recherche dans les carrières. Nous sommes plus réservés sur la perspective de prévoir l'évaluation éthique systématique des projets de recherche impliquant la personne humaine ne poursuivant pas de finalité biologique ou médicale. Une telle réforme nécessite un travail préparatoire pour être mise en oeuvre. Le Gouvernement souhaite par ailleurs attirer votre attention sur l'importance de prioriser les évolutions juridiques qui concernent les CPP, étant donné les multiples changements survenus récemment, lesquels sont longs à absorber pour des personnes exerçant leur activité de membre en sus de leur carrière professionnelle.

Comment garantir que les patients pourront être traités avec les produits les plus innovants, le plus tôt possible, et équitablement sur le territoire ? Comment anticiper l'arrivée de ces produits et assurer leur prise en charge, alors que les données, prometteuses, demeurent souvent précoces et ne permettent pas toujours une évaluation de droit commun ? Ces questions sont essentielles, et le Gouvernement s'est résolument engagé en faveur de dispositifs concrets pour apporter des solutions. La réforme de l'accès précoce relative aux médicaments, qui est entrée en vigueur en juillet dernier, a notamment permis de simplifier et d'accélérer les procédures dérogatoires, de systématiser la prise en charge immédiate des patients, de garantir un cadre d'éligibilité clair et d'assurer un maximum de prévisibilité aux entreprises sur le mode de financement. Ces évolutions ont produit des résultats très concrets. Ainsi, les patients français sont les premiers au monde à avoir bénéficié d'un traitement en prophylaxie, avec des anticorps monoclonaux actifs contre le variant omicron du virus SARS-CoV-2. Plus de 14 000 patients en profitent aujourd'hui, ce qui leur offre une meilleure protection, dans un cadre strict et sécurisé que nos autorités sanitaires ont fixé. Nous sommes, à date, le seul pays européen à proposer ce traitement. deuxième exemple est celui du traitement du cancer du sein métastasique sous une forme dite « triple négative ». Les patientes françaises en bénéficient depuis novembre 2021, ce qui fait de notre pays le premier en Europe à y donner accès.

En pleine tempête, le numérique en santé a montré qu'il était fondamentalement une solution efficace pour accéder aux soins et un allié de poids pour surmonter des contraintes inédites.

Cet espace numérique stocke tous les examens de santé : chaque patient peut renseigner ses antécédents, ses allergies et y classer ses ordonnances. J'invite chacun, ici et en dehors de cet hémicycle, à utiliser ce nouvel outil, dont les données sont évidemment sécurisées et hébergées en France.

de santé : plus de 2 milliards d'euros seront investis, dont 600 millions d'euros dans le seul secteur médico-social. Notre ambition est de moderniser, de sécuriser et de rendre interopérables les logiciels métiers dans les établissements et chez les professionnels de santé en ville, afin de fluidifier les échanges. Le troisième repose

En parallèle, l'utilisation des données à des fins de recherche, d'études ou d'évaluation s'est très fortement développée ces dernières années, ce dont on ne peut que se féliciter. Le système national des données de santé (SNDS) couvre intégralement l'utilisation des données en vie réelle, comme le démontrent les nombreuses études réalisées, que ce soit par la recherche académique, les agences ou les industriels du médicament. Nous comprenons que le développement du numérique en santé suscite